nous sommes réunis aujourd'hui, dans cet hémicycle, pour parler de l'avenir du sport français. Cet avenir, ce sont les jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024. Le Président de la République et le Premier ministre ont fixé un objectif clair et ambitieux. Pour réussir ce grand événement sportif, culturel et populaire, nous devons relever de multiples défis, bien sûr en termes de résultats sportifs, mais aussi d'association et d'implication de l'ensemble de nos concitoyens, notamment des jeunes, des femmes et plus largement de toutes celles et tous ceux qui sont éloignés de la pratique sportive, ainsi que de tous nos territoires, pas seulement Paris et la région Île-de-France. En ce sens, le label « Terre de Jeux » lancé par Paris 2024 est une formidable initiative visant à faire vivre les Jeux à travers toute la France et à en faire une magnifique fête populaire et fédératrice. Les cinq années qui nous séparent de 2024 sont par ailleurs une occasion unique de donner envie de sport à notre nation. Alors que, aujourd'hui encore, un Français sur deux ne pratique aucune activité physique, notre objectif est aussi d'augmenter le nombre de pratiquants dans notre pays. Du sport pour tous, quel que soit l'âge, les envies ou les aspirations de chacun. L'avenir du sport français, c'est également la réforme de notre modèle sportif, que je porte au sein du ministère des sports. En effet, j'ai pour ambition que ce nouveau modèle soit davantage au service de tous les Français et qu'il permette au sport d'occuper une autre place dans notre société. Avec l'accueil des Jeux, une nouvelle organisation doit être conçue pour perdurer bien au-delà de 2024 et permettre une transformation durable du sport en France. Le projet de loi, dont nous allons débattre cet après-midi, répond parfaitement à ces deux grands enjeux et permet de consacrer dans la loi des dispositifs structurels d'organisation qui ont été élaborés en lien étroit avec les acteurs du sport. Le premier dispositif prévu par le texte est celui des voies réservées à la « famille olympique » pour les Jeux de 2024. Conformément au cahier des charges du Comité international olympique, ces voies vont permettre aux athlètes, aux officiels, aux accompagnateurs, ainsi qu'aux véhicules de secours et de sécurité de circuler plus facilement. Grâce à la loi Olympique de mars 2018, le Gouvernement a pu insérer ce dispositif dans le cadre de l'ordonnance publiée le 20 mars dernier. C'est précisément cette ordonnance que l'article 1 du projet de loi ratifie, en nous permettant de respecter le délai qui nous était assigné. Toujours en complément de la loi Olympique, l'article 2 du projet de loi offre une garantie complémentaire de livrer, en temps et en heure, les infrastructures nouvelles construites pour les Jeux. Vous savez aussi bien que moi l'enjeu énorme que cela représente. Cet article acte ainsi une procédure exceptionnelle de règlement des litiges, puisqu'il désigne la cour administrative d'appel de Paris comme seule compétente. En cas de contentieux sur les décisions préfectorales prises en matière d'urbanisme, de construction ou d'aménagement en lien avec les Jeux, c'est elle qui statuera en premier et dernier ressort. En commission, ces dispositions ont été modifiées par plusieurs amendements. Afin de préserver les équilibres dégagés lors de l'élaboration de l'ordonnance, le Gouvernement souhaite revenir à la version initiale du texte s'agissant des voies olympiques comme des contentieux en matière de déférés préfectoraux. Au-delà de ces deux dispositions, qui s'inscrivent dans la continuité de la loi Olympique de 2018, je veux profiter de nos discussions pour rappeler que nous devons être au rendez-vous de ces Jeux, c'est-à-dire porter collectivement une politique publique ambitieuse en matière d'héritage. Cet héritage doit être à la fois durable, social et solidaire. Après une année 2018 consacrée à consolider le cadre juridique et financier des Jeux et lancer le programme de création des équipements, l'État et le COJO ont, dès 2019, mobilisé l'ensemble des territoires et engagé nos concitoyens dans le projet olympique. Cet héritage, c'est le fil conducteur de ma feuille de route. ma feuille de route. J'ai eu l'occasion de mettre en oeuvre cette feuille de route ces derniers mois par une série de plans d'actions concrets qui portaient sur différentes thématiques : la haute performance ; la recherche, au service de cette haute performance ; plus de sport à l'école et plus tôt dans la scolarité, avec par exemple le plan Aisance aquatique aquatique ; le sport-santé ; l'emploi sportif. J'aurai d'autres occasions de vous présenter ces actions. Cet héritage repose sur deux piliers : le développement de la pratique sportive ; le haut niveau et la haute performance.

J'ai souhaité que cette agence puisse être consacrée dans la loi, en y intégrant plusieurs garde-fous, qui ont été travaillés en étroite collaboration avec le Conseil d'État. C'est tout l'objet de l'article 3 du projet de loi qui nous occupe aujourd'hui. Constituée sous forme de groupement d'intérêt public, cette agence est chargée de favoriser le haut niveau et de développer l'accès à la pratique sportive. Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs qui y contribuent, partout sur les territoires. Le projet de loi rappelle ces principes et s'inscrit dans le cadre de la loi de 2011 sur les GIP. En complément, une convention constitutive signée par l'ensemble des membres fondateurs et approuvée par arrêté décrit plus largement l'objet, la composition et le fonctionnement précis de l'Agence. En préservant les équilibres entre les différentes parties prenantes, cette convention constitutive a permis de préciser le rôle de l'État. En particulier, celui-ci détient des droits de vote majorés en matière de haute performance, ainsi qu'un droit d'opposition sur les questions mettant en jeu les intérêts de l'État. En outre, à travers le ministre des sports, l'État a un pouvoir de proposition pour la nomination du président, du directeur général et du manager de la haute performance.

Plusieurs amendements adoptés en commission visaient à apporter des précisions au sujet de cette convention. Si je partage certaines de ces propositions, je ne souhaite pas pour autant que l'on en complexifie trop le processus d'élaboration. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter dans quelques instants. Je veux rapidement profiter des discussions qui nous rassemblent aujourd'hui pour lever quelques malentendus et confirmer devant vous que le ministère des sports continuera pleinement à jouer le rôle qui est le sien et à exercer les missions de nature régalienne en matière de contrôle, de sécurité et de régulation. Sur le reste de son champ d'action, le ministère se positionnera dans un rôle diffèrent, novateur et agile, dans une relation nouvelle avec les fédérations sportives et dans une plus grande ouverture vers l'ensemble des pratiques sportives. Le GIP que constitue l'Agence fera par ailleurs l'objet de différents contrôles, que le Gouvernement a souhaité renforcer dans le cadre de ce projet de loi, en le soumettant au contrôle d'un commissaire du Gouvernement, au contrôle économique et financier de l'État, ainsi qu'aux procédures liées à l'Agence française anticorruption. Il s'agit de garanties importantes que nous nous apprêtons à consacrer, aujourd'hui, dans la loi pour assurer, demain, le bon fonctionnement de l'Agence. Dans cet esprit et dans un objectif de transparence, le texte soumet le président du GIP, son directeur général et le responsable de la haute performance aux obligations relatives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Vos débats en commission ont également porté sur la présence des parlementaires au sein de l'Agence. Sachez que j'y suis favorable depuis le début. Je propose qu'ils puissent siéger au conseil d'administration de l'Agence au titre de personnalités qualifiées, comme cela était le cas au CNDS. Au-delà, il me paraît essentiel que les parlementaires puissent servir de relais à l'Agence ainsi qu'au ministère, notamment en faisant remonter les bonnes pratiques identifiées dans les territoires. La dimension territoriale de notre nouveau modèle sportif est un enjeu majeur. La question de son organisation territoriale doit naturellement être posée en cohérence avec le chantier gouvernemental en cours sur la réorganisation territoriale de l'État. À ce sujet, le projet de loi déposé par le Gouvernement confiait simplement au représentant de l'État dans les régions le rôle de délégué de l'Agence, notamment pour le plan financier. Ce volet territorial a été largement étoffé par vos travaux en commission. En particulier, deux dispositifs sur lesquels nous réfléchissons depuis plusieurs mois ont été intégrés au texte : d'une part, les conférences régionales du sport ; d'autre part, les conférences des financeurs. Si nous partageons pleinement le principe de ces propositions, le Gouvernement n'a néanmoins pas souhaité proposer d'amendements à ce stade, dans la mesure où des travaux sont en cours avec l'ensemble des membres du GIP pour préciser cette nouvelle organisation. J'ai naturellement demandé à ce que des parlementaires y soient associés et à ce que l'on puisse aboutir rapidement à un dispositif partagé, efficace et véritablement opérationnel. C'est la garantie d'une simplification de notre action au niveau local au bénéfice d'une plus grande proximité avec les associations et nos concitoyens. L'action du ministère des sports au niveau local repose pour beaucoup, vous le savez, sur le travail effectué avec engagement et professionnalisme, sur le terrain et au sein des fédérations, par les conseillers techniques sportifs. Vous connaissez aussi- j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'exprimer sur ce sujet lors de séances de questions au Gouvernement -le contexte de transformation, dans lequel nous sommes invités à redéfinir à redéfinir et à préciser la relation des CTS à l'État et aux fédérations sportives et, au-delà, leur action dans le cadre des politiques publiques mises en places. J'ai entendu la colère et les critiques émanant des premiers concernés. Je l'ai dit, et je le redis ici, je ne souhaite pas passer en force. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de nommer deux tiers de confiance, M. Yann Cucherat et M. Alain Resplandy-Bernard, qui sont chargés d'engager une large concertation, dans l'écoute et le dialogue. J'attends d'eux qu'ils formulent des propositions nouvelles en matière d'organisation structurelle du modèle, de portage des politiques publiques de haute performance et d'accès au sport pour tous Leur rapport me sera remis en octobre 2019. Dans cette attente, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, aucune réforme, aucun détachement, ne sera engagé, et le mouvement au titre de l'année 2019 est en train d'être mis en oeuvre. C'est pourquoi le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de la disposition adoptée en commission. Nous souhaitons laisser le temps à la concertation et permettre aux tiers de confiance de travailler sereinement.

Claude Kern, pour les échanges constructifs en amont de cette discussion en séance. Je sais votre attachement aux valeurs de l'olympisme et votre dévouement à faire des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 un grand succès sur tous les territoires. L'examen du présent projet de loi m'offre l'occasion de réaffirmer ma volonté de débattre avec vous et avec l'ensemble des parlementaires de l'évolution du modèle sportif français que je porte actuellement. Ce texte n'en est qu'une étape.

mais également en matière de développement de la pratique du sport pour le plus grand nombre, avec la volonté de lever un certain nombre de freins à celle-ci. Tout au long de ces démarches législatives, j'espère pouvoir compter sur votre soutien, comme la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a pu le faire, voilà quelques jours, en adoptant ce projet de loi. La parole

L'article 3 inscrit dans la loi l'Agence nationale du sport. Il ne s'agit pas d'une simple mesure technique visant à sécuriser juridiquement le statut de l'Agence, comme le laisse penser l'exposé des motifs. Cette reconnaissance législative constitue, en réalité, la pointe émergée d'un iceberg- le ministère des sports qui se détache malheureusement de plus en plus de l'État pour suivre sa propre route ... Toute la question est aujourd'hui de savoir où mènera cette évolution. La création de l'Agence nationale du sport ouvre en effet une nouvelle ère. Elle obligera le ministère des sports à se réinventer autour de ses missions régaliennes. Si sa pérennité semble garantie jusqu'à 2024, comme vous nous l'avez indiqué, madame la ministre, il ne fait guère de doute que son intégration progressive au sein au sein du ministère de l'éducation nationale- déjà envisagée au niveau des services déconcentrés -constitue un horizon probable, une fois que la flamme des Jeux de Paris se sera éteinte. Cette évolution du ministère des sports n'a pas fait l'objet d'un débat public. Le transfert obligatoire des CTS aux fédérations a été engagé de manière anodine, à travers un alinéa ajouté tardivement dans le projet de loi de transformation de la fonction publique, tandis que les deux plus importantes compétences du ministère des sports- la haute performance et le sport pour tous - lui sont enlevées à l'occasion du vote d'une disposition qui survient lors de l'examen d'un projet de loi portant ratification d'une ordonnance. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Je le dis avec d'autant plus de force que, au sein d'une commission comprenant de nombreux spécialistes du sport, nous sommes bien conscients des limites de notre modèle et de la nécessité de le faire évoluer. Je ne m'attarderai pas sur les conditions dans lesquelles nous avons préparé l'examen de ce texte- des conditions de travail loin d'être normalement confortables C'est pourquoi nous pensons qu'un débat sur les ambitions et les moyens que notre pays souhaite consacrer au sport est plus que nécessaire. Il n'est pas possible de découper par petits bouts le modèle sportif français en cherchant à faire le moins de bruit possible pour, en définitive, reporter le financement sur les collectivités territoriales, tout en essayant de maintenir la primauté de l'État. La recherche d'une gouvernance collégiale du sport demande du courage et de la sincérité. Or le statut de l'Agence nationale du sport vise à promouvoir la concertation entre les acteurs et la collégialité de la décision, tout en préservant une forme de primauté de l'État. Il suffit de regarder, par exemple, les droits de vote double pour l'État sur certains sujets, ou encore l'existence d'une convention d'objectifs permettant à ce dernier de définir la stratégie de l'Agence et le rôle de délégué territorial, confié au préfet de région. Le choix de confier la présidence de l'Agence au Délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques, ou Dijop, illustre également une certaine vision de la concertation. Si les mérites de cette nouvelle collégialité restent à démontrer, les nuages sont déjà nombreux à s'amonceler au-dessus de la nouvelle agence. Ses moyens financiers semblent inférieurs aux promesses initiales : ils sont plus proches des 300 millions d'euros que des 350 millions d'euros évoqués initialement. La disparition programmée des CTS fait planer une menace certaine sur la haute performance et, donc, sur la capacité de l'Agence à exercer sa mission, tandis que le devenir même de la structure n'est pas assuré au-delà des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Conseil d'État ayant indiqué que le choix du groupement d'intérêt public ne pouvait être que provisoire. Face à tant d'incertitudes, un débat démocratique était nécessaire. Nous ne pouvons donc que remercier le Conseil d'État d'avoir considéré que plusieurs dispositions de la convention constitutive de l'Agence nécessitaient de recourir à la loi, compte tenu, en particulier, des distances prises avec les règles relatives aux groupements d'intérêt public telles qu'elles ont été définies par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. L'examen au Parlement de l'article 3 ouvre la possibilité de dépasser les arguments de droit pour refonder notre politique sportive en apportant toutes les garanties nécessaires au Parlement, aux collectivités territoriales et au mouvement sportif. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons modifier et enrichir l'article 3, plutôt que de maintenir le comme le proposent certains de nos collègues. Supprimer l'article 3 reviendrait, en effet, à nier les insuffisances de notre modèle sportif, qui nourrit un fort mécontentement au sein des fédérations sportives comme des collectivités territoriales. Que dire, par ailleurs, de nos résultats sportifs, qui stagnent à un niveau souvent insuffisant compte tenu de la qualité de nos athlètes et des moyens mobilisés ? majorité, les membres de la commission considèrent donc utile d'accompagner cette réforme, qui a été conçue conjointement par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les fédérations sportives, tout en associant les acteurs du monde économique. Dans les premières esquisses de l'Agence, il était prévu que celle-ci se concentre sur le haut niveau dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce sont les acteurs de terrain qui ont souhaité que l'on n'oublie pas la pratique sportive. La double compétence est ainsi inscrite au fronton de l'Agence nationale du sport. Or cette double compétence est de plus en plus l'affaire des collectivités territoriales, lesquelles sont d'ailleurs de loin le premier financeur du sport pour tous. En outre, la décentralisation des Creps a fait des régions des acteurs incontournables de la haute performance. Voilà pourquoi il nous a semblé indispensable de préciser les modalités de la gouvernance territoriale de l'Agence nationale du sport. La seule précision à ce sujet que comportait l'article 3 du projet de loi concernait le préfet de région, qui se voyait reconnaître le rôle de délégué territorial de l'Agence. Cette désignation du préfet a suscité une réaction défavorable du mouvement sportif et des représentants des élus. Ceux-ci craignent, à la fois, un investissement variable de ce haut fonctionnaire selon les territoires et une gestion directive de la concertation, dans l'hypothèse où il lui reviendrait d'animer les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs. Pour répondre à ces inquiétudes, notre commission a souhaité circonscrire le rôle du délégué territorial et inscrire dès maintenant dans la loi le principe de la création des conférences régionales du sport en charge d'établir le projet territorial, ainsi que celle des conférences des financeurs. La rédaction de la commission prévoit que ces deux types de structures élisent leurs présidents en leur sein, ce qui exclut dans les faits une présidence imposée du préfet. J'ajoute que l'inscription des modalités de la gouvernance territoriale dans la loi permet également de mettre un terme au soupçon de report de la construction du second pilier de l'Agence nationale du sport relatif au développement de la pratique du sport. Je conclurai en évoquant l'avenir des CTS. Le Sénat a modifié l'alinéa 11 de l'article 28 du projet de loi de transformation de la fonction publique pour exclure un transfert obligatoire des CTS aux fédérations sportives. Pouvez-vous nous garantir, madame la ministre, que cette disposition, adoptée par le Sénat, sera maintenue dans le texte final ? Dans ce cas, nous pourrions renoncer à notre amendement à l'article 3, visant à donner mission au responsable de la haute performance de l'Agence de procéder à leurs affectations. Dans le cas contraire, il nous semblerait indispensable de préserver la possibilité d'une gestion coordonnée et dynamique de ce corps, indispensable à notre modèle sportif. un mot sur l'intitulé du projet de loi. Nous avons souhaité le modifier pour qu'il évoque la création de l'Agence nationale du sport. Cette mise en cohérence conforte l'importance de la réforme de notre modèle sportif initiée par ce projet de loi. La parole est à Mme

l'ordonnance prévoit que les voies de délestage des voies réservées, mais également celles qui peuvent être utiles, mais accessoires, seront déterminées, soit par le préfet de police en région Île-de-France,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Ouzoulias, pour la motion telle est la devise des olympiades de l'ère moderne. Votre projet de loi pourrait en être une brillante illustration, madame la ministre, tant il manifeste l'intention du Gouvernement d'aller plus vite dans la désagrégation du modèle sportif français, plus haut dans la transgression des droits du Parlement et plus fort dans sa volonté d'imposer cette réorganisation majeure sans aucune concertation. est bienveillant ! Tout commence lors de la discussion du projet de loi de finances pour l'année 2019 et le dépôt d'un amendement gouvernemental attribuant les taxes affectées au Centre national pour le développement du sport à une nouvelle Agence nationale du sport, sans existence. La rapporteure spéciale de ce budget pour l'Assemblée nationale avait exprimé alors ses plus vives réserves sur la transparence de cette manipulation budgétaire et, plus fondamentalement, sur l'opportunité de créer une nouvelle structure, à côté du Centre national pour le développement du sport et de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Dans le même esprit, le 29 novembre 2018, lors de l'examen du même projet de loi de finances, notre groupe, en la personne de notre collègue Pascal Savoldelli, s'était fermement opposé au transfèrement des crédits du Centre national pour le développement du sport vers un organisme dont le devenir, la gouvernance et les missions étaient encore indéfinis. Sans écouter les mises en garde et les critiques multiples, votre ministère a poursuivi dans l'improvisation en donnant, par un simple arrêté, le statut de groupement d'intérêt public à l'Agence nationale du sport. La fragilité juridique de ce dispositif vous oblige aujourd'hui à demander au Parlement de la doter d'une base légale un peu plus affermie, mais totalement dérogatoire.

Les bonnes pratiques législatives auraient dû vous conduire à nous présenter ce projet de réorganisation du sport de haut niveau dans une loi spécifique ou, à tout le moins, de nous expliquer sincèrement que c'était l'objet primordial du présent texte et que les articles de ratification n'y étaient rattachés que de façon accessoire. Nous regrettons vivement que vous n'ayez pas suivi l'injonction du Conseil d'État de faire apparaître dans le titre de ce projet de loi, de manière explicite, la création de l'Agence nationale du sport. À la demande de notre rapporteur, le sénateur Claude Kern, dont je salue le travail, notre commission a satisfait heureusement cette prescription. Mais il y a plus grave Dans son avis très critique, le Conseil d'État souligne que la nature juridique très particulière du groupement d'intérêt public, les missions générales qui lui ont été confiées par un arrêté et sa nécessaire pérennité imposent de lui octroyer, par la loi, un statut dérogatoire. Autrement dit, vous demandez au Parlement, par ce projet de loi, d'assurer l'existence juridique d'un organisme créé par un arrêté ministériel. La hiérarchie des normes en est renversée et le Parlement est sommé d'approuver une décision administrative constituée en fait accompli. Sa compétence est ainsi liée, ce qui est contraire au principe démocratique de la séparation des pouvoirs. C'est ce manquement qui motive le dépôt de la présente motion, conformément au troisième alinéa de l'article 44 de notre règlement. En février 2018, dans le champ de compétence de notre commission, le Gouvernement avait déjà procédé de la sorte en organisant par décret la plateforme Parcoursup et nous demandant ensuite d'assurer rétroactivement, par la loi, la solidité juridique de ces dispositions nouvelles. Déjà, il avait forcé notre décision en engageant une réforme d'ampleur, qui aurait compromis le bon déroulement de la rentrée si elle n'avait pas été confirmée par la loi. De la même façon, vous nous soumettez un projet de loi qui n'est que l'acte confirmatif d'un vaste projet de réorganisation du sport de haut niveau dont nous n'avons pas eu à connaître. En supprimant, par le décret du 20 avril 2019, le Centre national pour le développement du sport et en transférant ses ressources, ses biens et obligations à une nouvelle agence, dont le statut juridique est inapproprié pour poursuivre vous nous soumettez à un impératif fort peu respectueux des droits du Parlement et, singulièrement, de la liberté d'appréciation du Sénat. La loi du 29 octobre 1975, dite loi Mazeaud, fut l'un des outils essentiels de la construction du modèle sportif français. J'en rappelle les objectifs affirmés avec force dans son article 1 : « 1 : « Le développement de la pratique des activités physiques et sportives, élément fondamental de la culture, constitue une obligation nationale. [ ...] L'État est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive En liaison avec le mouvement sportif, l'État et les collectivités publiques favorisent la pratique des activités physiques et sportives par tous et à tous les niveaux [ ...]. » L'Insep, institué par son article 8, était chargé de l'encadrement du sport de haut niveau. Ses missions étaient alors de participer « à la recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et technique ; à la formation continue de niveau supérieur des personnels enseignants d'éducation physique et sportive, des conseillers techniques et des éducateurs sportifs et des éducateurs sportifs ainsi que des personnels des services de la jeunesse et des sports ; à l'entraînement des équipes nationales ainsi qu'à la promotion des sportifs de haut niveau. L'Agence nationale du sport, telle qu'elle est instituée par l'article 3 du présent projet de loi, semble recevoir dans ses dévolutions une grande partie de toutes ces missions, tant et si bien que monde sportif s'est interrogé sur la place qui serait laissée à l'Insep. Le Conseil d'État vous a expressément demandé dans son avis de préciser comment l'État, le Gouvernement et votre ministère continueraient de mettre en oeuvre les politiques publiques. Il vous a ainsi rappelé les obligations procédant de l'article 20 de la Constitution : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Afin de satisfaire cette obligation et de ne pas déposséder votre ministère de toutes ses capacités d'action, il vous a proposé de renforcer les moyens de contrôle de l'Agence par l'État et de mieux organiser ses moyens d'intervention en faveur des politiques publiques décidées par le Gouvernement. Le projet de loi transmis au Sénat a très peu été corrigé pour satisfaire ces demandes du Conseil d'État. C'est ce que vous avez appelé en préalable « travailler avec le Conseil d'État » d'État » ... Sur l'initiative de son rapporteur, dont je salue la valeureuse tentative de sauvetage, notre commission a considérablement amendé votre projet pour mieux définir le rôle et l'action de cette nouvelle agence, notamment dans les territoires. malgré ces propositions, il demeure légitime de se demander si la forme juridique du groupement d'intérêt public est appropriée pour répondre à ces objectifs ainsi redéfinis. Il serait plus judicieux de remettre en chantier la grande loi annoncée par votre prédécesseur, Mme Laura Flessel, lors de la présentation du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques, le 20 décembre 2017. Je la cite Je souhaite présenter début 2019 »- nous sommes en juillet -« devant le Parlement un projet de loi " sport et société " visant à encourager la pratique pour tous et partout, tout au long de la vie. Une loi pour le sport du quotidien, le sport plaisir, le sport santé, le sport éthique. Une loi qui parle aux gens. À ce texte et à sa préparation, je compte vous associer pleinement. Mes chers collègues, pour donner au Gouvernement la faculté d'honorer ses engagements, nous proposons au Sénat de surseoir à l'examen de ce texte en votant en faveur de la motion déposée par le groupe CRCE. Y a-t-il

la création de l'Agence nationale du sport est déjà effective depuis le 24 avril dernier. Cette entité constitue une pierre essentielle sur le chemin de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Refuser de discuter du présent projet de loi ne remettrait pas en cause le principe de son existence. En revanche, cela pourrait fragiliser juridiquement son statut et, ainsi, compliquer l'exercice de ses missions. ses missions. Il me semble donc préférable d'ouvrir au Sénat un débat, qui n'a pas véritablement eu lieu à ce jour, et de profiter de l'examen de ce texte pour apporter les garanties nécessaires aux collectivités territoriales et au mouvement sportif. L'avis est donc défavorable.

à l'unanimité dans cette enceinte, contrairement à l'Assemblée nationale. On ne peut pas se dédouaner de la nécessité de créer les bonnes conditions pour la tenue des jeux Olympiques de 2024

Pendant plus d'un mois, nous vous avons demandé de venir devant la commission, comme le fait tout ministre pour défendre son texte, l'expliquer, dialoguer avec les parlementaires, essayer de l'enrichir, de l'améliorer. C'est le travail normal que nous faisons avec tous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

du scrutin n° 159 : Le Sénat n'a pas adopté. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Claude Malhuret.

Les jeux Olympiques et Paralympiques offrent des moments uniques de communion universelle, pendant lesquels des milliards d'hommes et de femmes aux quatre coins du globe vibrent ensemble aux exploits de leurs champions. Autant dire que l'échéance nous oblige. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui doit permettre à la France d'être à la hauteur de l'enjeu. Pour la deuxième fois, le Parlement est appelé à voter des dispositions spécifiques pour doter la puissance publique des outils adaptés. C'est notamment l'objectif des deux premiers articles, l'un ratifiant l'ordonnance relative aux voies réservées et à la police de la circulation, l'autre attribuant à la cour administrative d'appel de Paris les contentieux de déférés préfectoraux portant sur des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière. Ces deux articles découlent essentiellement de décisions déjà actées par le Parlement et n'appellent pas, de ce fait, de commentaire particulier. Mais, contrairement à ce qu'indiquait l'intitulé initial du projet de loi, le texte dont nous discutons aujourd'hui ne se réduit pas pour autant à de simples mesures techniques et opérationnelles. Il a une portée politique, que les travaux de la commission ont clairement exposée. « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde », disait Camus. Il faut donc saluer l'initiative de notre collègue et rapporteur Claude Kern, qui a proposé de renommer le projet de loi afin de lui donner un titre qui correspond mieux à la réalité et sans doute, ce faisant, de diminuer le malheur de ce monde. En effet, le texte ne vise pas seulement la ratification d'ordonnances. Il régularise l'existence de l'Agence nationale du sport, dont le principe avait déjà été acté. Compte tenu des missions que vous souhaitez lui confier, madame la ministre, il apparaît nécessaire d'avoir un débat en bonne et due forme sur les implications de ces décisions pour notre modèle sportif. La méthode que vous avez retenue pour soumettre ce projet de loi peut sembler un peu cavalière, notamment dans la succession des décisions, d'abord réglementaires, puis législatives, ou encore en ce qui concerne le temps d'échange et de débat en commission. Je n'insisterai pas sur ce sujet : Mme la présidente de la Ce projet de loi a pour objet, non seulement la bonne organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, mais aussi la réorganisation du modèle sportif de la France. Avec la création de l'Agence nationale du sport, c'est bien de l'avenir de la pratique sportive en France qu'il est question, tant pour les amateurs que pour les professionnels. Ce changement d'approche constitue une décision politique au sens fort du terme. C'est pourquoi j'approuve la proposition de la commission d'associer des députés et des sénateurs à la gouvernance de l'Agence et de soumettre sa gestion au contrôle du Parlement, qui a toute légitimité pour prendre part au pilotage de cette institution. Mais la réorganisation du modèle sportif français concerne au premier chef les collectivités territoriales. Elles doivent prendre toute leur part dans ce dispositif ; le présent texte en pose le cadre et fixe les objectifs. Elles sont les acteurs les plus indiqués pour animer la pratique sportive dans nos territoires, à proximité immédiate de nos concitoyens. Les aménagements introduits en commission, notamment concernant le principe d'une gouvernance territoriale de l'Agence nationale du sport, me semblent à cet égard tout à fait pertinents. Ils doivent contribuer à ancrer la politique nationale du sport dans les territoires. En effet, le sport est un puissant vecteur d'intégration sociale. On y apprend à respecter l'autre pour ce qu'il fait, indépendamment de ce qu'il est. Camus, encore lui, disait que ce qu'il savait de plus sûr en matière de morale, il l'avait appris dans un stade de football. Je ne sais si j'ai raison de citer cette phrase : le football de l'époque de Camus n'a pas grand-chose à voir parce qu'il renforce le lien social, parce qu'il donne sa chance à tous, parce qu'il favorise toujours celui qui s'efforce et persévère, le sport est une école de la République, dans les villes comme dans les campagnes, pour chacun et pour chacune. Nous aurions bien tort de nous en priver. Parce que le sport est si utile à la cohésion sociale, la puissance publique doit favoriser les conditions de sa pratique par toutes et par tous. Mais parce que le sport est aussi utile en matière de diplomatie internationale, par l'influence qu'il exerce par-delà les frontières, la puissance publique doit également créer les conditions propices à l'émergence de nouveaux talents et de futurs champions qui, avant d'aller décrocher l'or olympique, commenceront par s'entraîner là d'où ils viennent. pour la politique du sport comme pour bien d'autres domaines, un modèle centralisé et étatique se révèle bien souvent moins efficace et moins inclusif qu'un modèle décentralisé et collégial. Il s'agit, dans ce cas comme dans d'autres, de faire confiance aux acteurs de terrain plutôt qu'aux technocrates éloignés du terrain. Le groupe Les Indépendants votera donc le projet de loi tel qu'amendé par la commission, afin de soutenir le renouvellement du modèle sportif français

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme cela a été rappelé, nous nous retrouvons pour la deuxième fois dans cet hémicycle pour examiner des dispositions législatives qui doivent permettre à la France de faire des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 une grande réussite. Disons-le d'emblée, madame la ministre : le Sénat adhère au but fixé par ces textes, car nous sommes tous conscients que, derrière l'organisation de cet événement sans précédent, c'est l'image de la France dans le monde qui sera en jeu. pour réussir, nous devrons relever un double défi. Le premier défi est financier. Chacun a en mémoire les dérives financières qui ont secoué les précédentes éditions- je sais ce dont je parle, car Rio est voisin de la Guyane. Il est donc primordial que la France soit à la hauteur de l'enjeu et maîtrise les coûts annoncés. Le second défi est plus profond. Il réside dans notre capacité à valoriser l'olympisme par-delà l'événement lui-même, par-delà l'élan d'enthousiasme sportif qu'il suscitera jusqu'à ce que la flamme soit éteinte. À cet égard, l'olympiade culturelle qui précédera de quatre ans l'ouverture des Jeux est un très bon outil.

Cela étant dit, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'examen d'un texte pour le moins singulier. En effet, d'abord conçu de manière purement technique, ce projet de loi a rapidement évolué face à la nécessité posée par le Conseil d'État de passer par la loi pour créer l'Agence nationale du sport. Tout d'abord, il nous est proposé, avec deux premiers articles bienvenus, la ratification de l'ordonnance relative aux voies réservées à la circulation de certains véhicules et à la police de la circulation. Si l'on pouvait légitimement penser que ces mesures concernaient davantage le domaine réglementaire, le recours à la loi était toutefois nécessaire. En effet, la répartition des compétences, s'agissant de la police de la circulation, relève directement du pouvoir normatif. La perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est donc une chance à saisir pour faire évoluer le modèle sportif français, régulièrement mis à l'index. Celui-ci doit être en phase avec les nouvelles attentes des pratiquants et des acteurs sportifs représentés dans toute leur diversité et, plus largement, avec les enjeux de notre société. Aussi l'article 3 vient-il préciser l'Agence nationale du sport sous la forme d'un groupement d'intérêt public, ou GIP, dont l'objectif est précisément de renforcer les capacités sportives du pays sur le fondement d'une gouvernance collégiale et concertée. Le principe ne pose aucun souci majeur. Au contraire, notre rapporteur a lui-même souligné la pertinence du recours au GIP, en ce qu'il permet une souplesse de gestion et de financement. Pour autant, reconnaissons-le, il il est quelque peu frustrant pour les parlementaires que nous sommes d'effleurer ainsi l'Agence nationale du sport sans évoquer davantage son organisation, son mode de gouvernance ou encore sa pérennité. Le sujet n'est pas anecdotique. Comme l'observe le Conseil d'État, la création de cette nouvelle agence revient pour l'État à se dessaisir des principales dimensions de la politique du sport le soutien au sport de haut niveau et à la haute performance, d'une part, le développement de l'accès à la pratique sportive, d'autre part. C'est la raison pour laquelle notre rapporteur, que je salue de nouveau pour son travail, a souhaité profiter de ce texte pour ouvrir le champ de notre débat. Je me réjouis personnellement de l'occasion qui nous est donnée de parler de sport, tant les débats techniques autour des JO 2024 peuvent parfois se révéler frustrants. Dans le détail, notre commission a voulu préciser la gouvernance, l'organisation territoriale et les moyens de cette nouvelle agence. Les membres de notre groupe soutiennent les modifications opérées en faveur d'un rôle accru des parlementaires dans la politique sportive de la France. Il semble en effet important que certaines commissions puissent donner un avis sur la convention d'objectifs. Ils portent également un regard bienveillant sur le recentrage du rôle du préfet de région comme délégué territorial ainsi que sur la création d'une conférence régionale du sport. nous sommes opposés à la décision de confier au responsable de la haute performance de l'Agence l'affectation et l'évaluation des conseillers techniques sportifs dans les fédérations agréées. Si j'ai personnellement soutenu la position récente de notre commission contre un transfert obligatoire des CTS aux fédérations sportives, c'est précisément parce qu'un temps de concertation me paraît indispensable. Aussi, il me semble tout autant précipité de confier la gestion des CTS à l'Agence nationale du sport, tout juste créée. Je note d'ailleurs que le collectif des 1 300 CTS comme l'association des directeurs techniques nationaux n'y sont eux-mêmes pas favorables. Madame la ministre, je vous sais pleinement investie pour faire évoluer le modèle sportif français ; un modèle en vertu duquel l'État est partenaire auprès des acteurs responsables et engagés que sont les fédérations, les collectivités et le monde de l'entreprise. Aussi, je ne doute pas que vous saurez nous rassurer pour poser ensemble la première pierre d'un débat plus large ; un grand débat que nous aurons en 2020, je l'espère, autour du projet de loi Sport, texte qui vous est cher et que nous appelons tous de nos voeux. Pour l'heure, notre groupe votera le présent projet de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, qui nous est présenté bien souvent comme un texte technique, est en réalité lourd de conséquences pour l'organisation de notre modèle sportif- nous avons déjà abordé le coeur de ce projet de loi, c'est évidemment la création de l'Agence nationale du sport, contrairement à ce que son titre laissait entendre. Madame la ministre, cette méthode ne fait pas honneur à votre ministère. Il aurait été plus opportun de conduire un large débat sur notre modèle sportif, sur ses atouts, sur ses défauts et sur les éventuelles modifications à lui apporter, avant de définir les structures et les outils nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique sportive. De ce point de vue, vous garantissez un projet de loi d'ampleur sur le sport d'ici à 2020, mais le Premier ministre n'en a pas dit mot dans son récent discours de politique générale, ce qui n'est pas pour nous rassurer. sans attendre cet hypothétique débat, vous réformez profondément le modèle sportif français par la création, que vous demandez au Parlement de ratifier, d'une d'une agence dont les missions consacrent une nouvelle séparation en France entre le sport de haut niveau- la haute performance -et le sport de masse. Or tous les acteurs de terrain le savent : il est absurde et vain de vouloir l'un sans l'autre. C'est là importer une vision étrangère, anglo-américaine pour être précise, sur laquelle notre culture nationale, totalement différente, ne peut se calquer, et qui est d'ailleurs loin de tenir toutes ses promesses dans les pays où elle s'applique, même en prenant en considération les seuls critères du sport de haut niveau. Plus grave encore : cette agence, à laquelle vous nous demandez, pour la forme, de donner notre assentiment, marque un désengagement inédit de l'État et ouvre la porte à une privatisation du sport, qui rompt avec tout ce qu'est le modèle français du sport. Ainsi le monde économique aura-t-il son mot à dire sur la politique du sport et l'utilisation des deniers publics en matière sportive. On se demande bien au nom de quoi l'État se dessaisirait volontairement de ses prérogatives au profit d'un groupement d'intérêt public tout en continuant à le financer. C'est le contraire qu'il faudrait faire : désintoxiquer le sport, tout au moins certaines disciplines, de l'argent, qui conduit parfois aux antipodes des valeurs de l'olympisme. En revanche, dans d'autres disciplines, dans le sport amateur, et ce dans nombre de nos territoires, on tire le diable par la queue, si vous me permettez l'expression.

indique que l'Agence nationale du sport déploiera son action au niveau régional les Creps, pour ce qui concerne le sport de haut niveau, Creps dont la voilure- doit-on le rappeler ? -a été amputée d'un tiers et qui, aujourd'hui, reposent essentiellement sur les régions. Mais c'est les directions académiques des services de l'éducation nationale que s'organiserait le sport pour tous, en même temps que le préfet serait le délégué territorial de l'Agence. Et il faut ajouter la création d'un délégué auprès du recteur de région académique pour animer le réseau des équipes chargées de ses missions. Ministère, Agence nationale du sport, Creps, Dasen, préfet, recteur, sans même parler des modifications impliquées par le service national universel concernant le sport : nos un bon sens de l'orientation pour trouver le bon interlocuteur et, ainsi, mener à bien les projets sportifs dans leur commune ou leur bassin de vie ! Ce que vous nous proposez n'est donc pas davantage justifié par un besoin de simplification que par le projet de fond qui le sous-tend et on voit difficilement ce que le pays, les élus comme les citoyens, a à gagner dans tout cela., ce que nous y perdrions est assez clair. La logique globale, c'est la mise en cause de l'existence même d'un véritable ministère des sports. Le travail de sape a déjà commencé, comme en témoigne la baisse du budget du sport de 6 % cette année, après une baisse de 7 % l'année précédente. Le sort réservé aux CTS est, dans ce cadre, tragiquement parlant : le Gouvernement veut transférer un CTS sur deux vers les fédérations sportives et supprimer le concours, ce qui conduirait de fait à l'extinction, à moyen terme, de ce corps. Mes chers collègues, je crains que nous ne perdions le point marqué ensemble, ici, la semaine dernière, en excluant les CTS des détachements d'office projet de loi sur la fonction publique, si nous décidions de les transférer à l'Agence nationale du sport. Puisqu'une pause dans ces transferts a été obtenue- madame la ministre, puisque la mission Cucherat Resplandy-Bernard doit rendre ses conclusions au mois d'octobre prochain- vous l'avez également rappelé -, n'optons pas pour un remède qui pourrait se révéler pire que le mal. Le sport, en France, c'est bien davantage que le sport. Dans beaucoup de nos territoires, une partie essentielle de la cohésion sociale s'y joue. le plan national, de grands événements jouent un rôle fédérateur, de cohésion nationale, à l'image du soutien populaire qui s'est tout récemment exprimé à l'égard de notre équipe féminine de foot. C'est aussi, au quotidien, un vecteur d'engagement pour des milliers de bénévoles qui font vivre le sport de proximité, dans presque toutes nos communes. Déstabiliser ce modèle sans même avoir conduit un débat de fond sur les orientations en matière de politique sportive, alors que le haut niveau se prépare pour les prochains jeux Olympiques et Paralympiques et que la France elle-même se prépare à accueillir les JO de 2024 ; déstabiliser ce modèle, qui repose sur l'engagement de plus en plus fragile de ces millions de bénévoles, est extrêmement risqué. Nous voudrions vous en convaincre, madame la ministre ! La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, par ses articles 1 et 2, le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui porte ratification de l'ordonnance du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En outre, il porte dérogation aux dispositions de droit commun s'appliquant aux contentieux des déférés préfectoraux devant les tribunaux administratifs. Je ne m'appesantirai pas sur ces deux articles, portant application de la loi du 26 mars 2018. Mon intervention se concentrera sur l'article 3, qui vient avaliser la création, déjà effective, de l'Agence nationale du sport. Fallait-il appréhender la refonte du modèle sportif français par un texte de circonstance, par un seul article, en procédure accélérée, d'un projet de loi visant à sécuriser juridiquement l'Agence nationale du sport à la demande du Conseil d'État ? Ou bien fallait-il fixer législativement le cadre d'une politique sportive nationale, à l'intérieur duquel l'Agence serait appelée à jouer, ou non, un rôle d'opérateur ? Le moment n'était-il pas venu de réinterroger les notions de missions de service public, de délégation ou encore d'agrément, le sport et la société de 2019 n'étant pas le sport et la société de 1984 ou de 2000 ? Je fais bien sûr référence à la loi du 16 juillet 1984, dite Avice, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, corrigée par la loi dite Buffet du 6 juillet 2000. Raccrocher la problématique de l'Agence, créée en avril dernier, aux questions de voies réservées et de police de la circulation inhérentes aux JO de 2024 n'est-il pas pour le moins cavalier ? Fallait-il inviter les parlementaires à cette importante phase de consultation de 2018 sur la gouvernance du sport, consultation sous-jacente à la mise en oeuvre de l'Agence Fallait-il limiter la réforme du modèle sportif à une mutation du CNDS, par une modification de ses règles statutaires et l'élargissement de son mode de gouvernance, ou bien aller plus loin ? Fallait-il faire le choix de la forme juridique du GIP, d'un établissement public à caractère administratif, voire d'un établissement public à caractère industriel et commercial ? Fallait-il commencer par installer une agence ayant comme objet la haute performance, en reprenant la formule de Tony Estanguet- isoler le haut niveau, en mode commando » -, avant, éventuellement, de l'élargir au développement des pratiques ? Ou bien fallait-il, dès le départ, tenter de relever les deux défis Je pose beaucoup de questions et reste muet sur les réponses. Pourquoi ? Tout simplement parce que le texte dont nous sommes saisis ne nous sollicite pas sur ces questions majeures ! Pourtant, le cap fixé par l'Agence ne saurait résulter d'une confusion entre les fins et les moyens. Il importe de créer les conditions pour que se déploie une bonne combinaison entre les politiques sportives territoriales et les plans de développement des fédérations. Ne pas réunir ces conditions compromettrait l'atteinte des ambitions affichées : 80 médailles aux JO de 2024 et 3 millions de pratiquants supplémentaires.

Rappelons que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, et alors que cette instance n'avait aucune existence juridique, un amendement gouvernemental a désigné « l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement à l'accès à la pratique sportive » comme affectataire, au plus tard le 1 septembre 2019, des financements jusque-là versés au Centre national pour le développement du sport. Cette annonce posait immédiatement la question du respect des engagements financiers en cours et suscitait l'inquiétude des collectivités territoriales pour le financement et la pérennité de leurs projets.

Aujourd'hui encore, la demande sociale transcende largement, et de plus en plus, les disciplines olympiques- certains évoquent une « ubérisation » du sport -avec les activités hors structures, moins élitistes, parfois activités physiques de pleine nature, parfois activités d'essence très urbaine. Ainsi l'offre du service public doit-elle dépasser la seule pratique sportive et prendre en compte les expressions corporelles nouvelles. L'article 3 ne fait pas référence à la dimension budgétaire de l'Agence, la traduction administrative du projet de politique sportive s'est toujours heurtée, en France, au manque de moyens. Quand une organisation nouvelle se met en place- c'est le cas ici -, elle implique une nouvelle économie qui devra faire ses preuves. Une dynamique de financement est donc attendue, créée par une coopération harmonieuse des quatre acteurs impliqués, sans sous-estimer la faiblesse actuelle du mécénat d'entreprise et les difficultés financières des collectivités territoriales. Le succès de la démarche sera évalué à l'aune de la mobilisation de nouvelles ressources. Je rappelle que les moyens affectés au CNDS ont chuté de moitié depuis deux exercices budgétaires, passant de 260 millions d'euros à 131,4 millions d'euros entre 2017 et 2019. Cette large diminution des ressources est directement liée au plafonnement de la part du produit de deux des trois taxes affectées alimentant son budget, ainsi qu'à la suspension, depuis 2018, du prélèvement exceptionnel supplémentaire de 0,3 % sur les gains de la Française des jeux, permettait de dégager 25 millions d'euros chaque année. Je me permets un clin d'oeil : 25 millions d'euros, c'est exactement le montant nécessaire pour expérimenter le pass sport de 500 euros pour 50 000 bénéficiaires ! Aujourd'hui, le sport n'est plus seulement du sport, tant il est évident que des facteurs qui lui sont extérieurs ont investi son domaine propre, au point parfois de le dénaturer. Le sport est nu ; il ne recèle aucune vertu propre. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Michel Serres écrivait : « Instrument pédagogique hors pair, le sport interdit le mensonge, le sport apprend le réel. Mais maintenant, s'il ne s'agit que de gagner, alors je suis écoeuré jusqu'à la mort. » Aussi sommes-nous très attachés à l'efficacité que nous sommes en droit d'attendre de l'État dans l'affirmation de la mise en oeuvre d'une vision éthique du sport, par-delà le simple énoncé des valeurs dont tout le monde se gargarise et que chacun conjugue à sa propre sauce. L'histoire est là pour nous rappeler que c'est au nom des grands principes que les pires dérives cherchent leurs justifications : nationalisme, tricheries, manipulation de compétitions, corruption, dopage, violence, alors que le sport est d'abord un humanisme. Puisque l'Agence devient la pierre angulaire du sport de la République, il faudra préciser ses missions en matière d'exploitation optimale des vertus et des apports des APS, et dans tous les domaines sport et éducation, sport et entreprise, sport et emploi, sport et aménagement du territoire, sport et tourisme, sport et insertion sociale, sport et lutte contre toutes formes de discrimination, sport et développement durable, Considérant que notre efficacité de parlementaires, dans les missions d'évaluation et de contrôle qui nous sont confiées, est renforcée lorsque nous sommes pleinement intégrés au sein des différentes structures, je défendrai un amendement prévoyant d'ajouter dans les statuts de l'Agence la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de son Par ailleurs, veillons à ne pas démotiver les bénévoles sur le terrain, qui trouvent souvent le plein accomplissement de leur engagement dans un fonctionnement harmonieux avec les professionnels de l'encadrement. J'ai à l'esprit, bien évidemment, le rôle des conseillers techniques sportifs, dont la situation doit être traitée avec diplomatie et avec un réalisme à la hauteur de l'irremplaçable service qu'ils rendent depuis des décennies au sport français. Sans les bénévoles, les encadrants et les supporters, que serait le club, cellule de base de toute l'architecture ? L'État doit aussi faire naître et encourager les bonnes volontés qui acceptent d'animer et de diriger les cellules sportives et les aider dans leur action. J'ai déposé un amendement de suppression de l'alinéa de l'article 3 qui vise à faire de l'Agence, à travers son responsable de la haute performance, le gestionnaire des CTS, tant il me paraît évident qu'un GIP n'a pas à exercer la direction des

l'ANDES ne cesse de répéter, fort justement, que 22 % des installations sportives ont plus de cinquante ans d'âge et nécessitent une rénovation. Tout attendre d'une instance nouvelle, seulement parce qu'elle installerait autour de la table ces quatre composantes, serait illusoire. Il faudra, dans le cadre des dispositifs décentralisés envisagés, des diagnostics partagés, des acteurs volontaires, des choix assumés, des contractualisations et des budgets respectés, une osmose entre sport de performance et sport du quotidien. Oui, madame la ministre, au-delà des observations que je viens de faire, le temps d'une refondation du sport est venu, vous le dites vous-même ! Une loi en sera le passage obligé. on ne saurait prendre le risque de s'orienter vers une disparition du sport considéré comme un service public. Je note d'ailleurs que la fameuse agence britannique UK Sport, qui semble susciter beaucoup de fantasmes chez nous, est placée sous la tutelle du ministère de la culture, des médias et du sport, mais avec un fonctionnement totalement autonome.

Le projet de loi en discussion ce jour nous avait été présenté par le Gouvernement comme un texte technique, il est pourtant bien plus que cela ! Il représente aujourd'hui pour nous, avant tout, l'opportunité précieuse d'ouvrir un débat le Parlement sur un sujet majeur auquel celui-ci n'avait jusqu'ici pas été associé : l'avenir de la politique du sport en France, de son ministère et la création de l'Agence nationale du sport. Nous saluons l'initiative de notre rapporteur, Claude Kern, qui a replacé l'examen de ce projet de loi dans une perspective cohérente avec la réalité des enjeux qui sont devant nous.

Cette nouvelle collégialité dans la conduite d'une politique publique marque une rupture culturelle significative : comme l'a voulu le Conseil national de la Résistance, c'est l'État, et lui seul, qui demeure en France, depuis soixante-quinze ans, le garant de l'intérêt général. Les acteurs du sport et les collectivités territoriales ont appelé de leurs voeux une évolution du modèle sportif français, ils se sont impliqués dans la réforme en cours, nous ne l'ignorons pas. que nous voulons le débat, nous ne souscrirons pas à la proposition de suppression de l'article 3, même si les insuffisances de ce texte sont nombreuses. L'exécutif affiche sa volonté, à travers la création de cette nouvelle agence, de favoriser le dialogue et la concertation sur le terrain, tout en conservant une forme de primauté de l'État. Les travaux de notre rapporteur pointent pourtant le caractère pour le moins précaire d'un tel équilibre.

La proposition de notre rapporteur de prévoir la présence de parlementaires au sein de l'Agence nationale du sport permettra ainsi, très opportunément, à la chambre haute et à la chambre basse d'exercer leur pouvoir de contrôle. Dans la même perspective, la faculté donnée aux commissions des affaires culturelles et à celles des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale de formuler un avis sur les conventions d'objectifs signées entre l'État et l'ANS, ou encore de suivre leur mise en oeuvre, manifeste notre volonté de veiller à la pérennité d'un service public du sport en France. La capacité de l'ANS à remplir efficacement ses missions demeure aussi suspendue au sort qui sera réservé aux conseillers techniques sportifs.

d'abord, pour les premiers intéressés, mais également pour l'ensemble du sport de haut niveau français, et ce alors que la France s'apprête à accueillir les Jeux de la trente-troisième olympiade de l'ère moderne. Soucieux d'apporter des éléments de réponse à la situation actuelle, notre rapporteur souhaite faire affecter les conseillers techniques sportifs par le responsable de la haute performance à l'ANS.

qui ignorent encore tout de l'organisation territoriale de l'Agence. En choisissant d'inscrire d'ores et déjà dans la loi les principes de sa gouvernance territoriale, notre rapporteur fait oeuvre utile, l'absence de calendrier de déploiement de son volet territorial fait en effet craindre aux acteurs locaux la mise en place, d'ici à 2024, d'un dispositif transitoire privilégiant le très haut niveau. Telle n'était pourtant pas leur attente.

Les inquiétudes autour des moyens financiers dévolus à l'ANS sont également vives. Le compte risque de ne pas y être. Les ressources allouées au sport en France ne devraient pas sortir intactes de ces bouleversements en matière de gouvernance, qui, comme bien souvent, ont également une motivation budgétaire. Comme l'a justement relevé le Conseil d'État, la création de l'ANS est lourde de conséquences. Elle conduira l'État à se dessaisir des deux principales dimensions de la politique du sport en France : le soutien au sport de haut niveau et à la haute performance sportive que le développement de l'accès à la pratique sportive. Le Gouvernement ayant privilégié la voie réglementaire pour créer l'Agence, le Parlement n'avait pas eu la faculté de débattre de cette réforme, laquelle est tout sauf anecdotique. Le groupe du RDSE se félicite donc que la Haute Assemblée ait pu oeuvrer sur ce sujet et entreprendre d'apporter des éléments de réponse aux nombreux points encore en suspens. Notre groupe formulera également des propositions au cours du débat, afin, notamment, d'affirmer le rôle des élus locaux et d'ancrer l'Agence dans la proximité. Comme le disait le baron de Coubertin, l'important, c'est de participer mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer, dans la tribune d'honneur du Sénat, une délégation de quatre députés membres du groupe d'amitié Corée du Sud-France de l'Assemblée nationale de Corée du Sud, conduite par M. Sye kyun Chung, président du groupe d'amitié et ancien président de l'Assemblée nationale Ils sont accompagnés par notre collègue Mme Catherine Dumas, présidente du groupe d'amitié France-Corée du Sud. La délégation est en France jusqu'au 4 juillet, pour une visite d'étude consacrée, notamment, au développement durable. Elle s'est rendue hier sur le site de recherche et d'innovation de Samsung France et a rencontré aujourd'hui plusieurs de nos collègues, en particulier MM. Philipe Dallier, premier vice-président, et Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, à nos homologues de l'Assemblée nationale sud-coréenne, la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour.

nul n'aurait pu penser qu'il soulèverait un débat aussi structurel sur l'avenir du sport dans notre pays. De fait, l'essentiel de nos discussions, en commission et ici même en séance, ainsi que de nos amendements, ne porte pas sur les voies réservées et la police de circulation pour les jeux Olympiques de 2024. Loin de moi l'idée de minimiser les enjeux que recouvrent les deux articles qui abordent ce sujet, nos estimés rapporteurs, que je remercie pour la qualité de leurs travaux, les ont d'ailleurs fort bien mis en avant dans leurs rapports. Ainsi, ce ne sont pas moins de 360 kilomètres de voies routières qui devraient être réservés

Si nous en comprenons cependant la nécessité, nous soutenons les amendements d'encadrement et de précision introduits par notre collègue Muriel Jourda, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je ne peux toutefois m'empêcher de noter que cette ordonnance intervient dans un contexte de retard important des différents grands projets d'infrastructures censés désengorger la région capitale et fluidifier les déplacements, notamment de banlieue à banlieue. à l'esprit le Grand Paris Express, dont même les lignes desservant le village et les sites olympiques risquent de ne pas être prêtes, ou encore le Charles-de-Gaulle Express. Le représentant des Yvelines que je suis déplore également fortement que la ligne 18 n'ait pas été jugée prioritaire alors que pas moins d'une dizaine de compétitions auront pour cadre ce département. Certes, le Gouvernement ne saurait être tenu pour seul responsable du retard de projets lancés bien avant son arrivée aux responsabilités. si la mise en place dans les délais annoncés de ces infrastructures ferroviaires n'aurait pas rendu inutile la réservation de voies de circulation, elle en aurait sans doute atténué les effets sur la fluidité de la circulation automobile, notamment pour leurs usagers quotidiens. Comme je le disais, l'essentiel de ce projet de loi n'est pourtant pas là. Comme l'a souligné notre rapporteur Claude Kern, l'article 3, traitant de l'Agence nationale du sport, n'était, en effet, pas prévu à l'origine par le Gouvernement. Il a été ajouté par souci de sécurité juridique, laissant penser, au premier abord, à quelques mesures techniques ne méritant pas que nous nous y attardions, à tel point qu'il n'a pas été jugé utile de le mentionner dans le titre du projet de loi. loi. Fort heureusement, nous nous y sommes intéressés, car les mesures que contient cet article sont de nature à déterminer l'avenir de l'ensemble du monde sportif français : elles traitent des modalités de mise en place de l'Agence nationale du sport, dont la création avait déjà été entourée d'un relatif flou artistique. Le Gouvernement justifie le choix de créer l'Agence nationale du sport sous la forme d'un groupement d'intérêt public, un GIP, par le contexte particulier de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques par la France en 2024. Si cette forme juridique a été jugée préférable à celle d'un établissement public, en raison, notamment, selon l'étude d'impact, de la collégialité renforcée qu'elle autorise et de la plus grande souplesse de fonctionnement qu'elle permet, le Conseil d'État relève que, sur plusieurs points, ce GIP s'écarte du régime général de ces groupements, ce qui conduit à s'interroger sur la véritable nature juridique de l'Agence. Le Conseil d'État considère, en outre, que le choix du statut de GIP n'est adapté qu'à des collaborations dédiées à un projet ou à la phase de mise en place d'une agence. Pour ces raisons, il estime que cette structure, créée pour des raisons très circonstancielles, n'a pas vocation à demeurer pérenne dans la forme initiale dessinée par le projet de loi. Nous nous interrogeons donc sur la démarche du Gouvernement, à nous soumettre des dispositions sur lesquelles la réflexion mériterait, manifestement, d'être approfondie. Il est regrettable à ce titre, madame la ministre, ainsi que l'a souligné la présidente Catherine Morin-Desailly, que vous ne soyez pas venue en débattre avec nous lors de nos travaux en commission.

Par ailleurs, nous déplorons que les collectivités territoriales ne soient pas mentionnées dans le projet de loi. Nous soutiendrons donc les amendements de notre rapporteur Claude Kern allant dans le sens de leur pleine intégration dans le nouveau dispositif.

Comme bon nombre d'entre nous, en lisant « Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 je m'attendais à un texte technique et, si possible, pragmatique, visant simplement à faciliter l'accès aux sites olympiques. Nous savons bien, désormais, que les intentions du Gouvernement sont tout autres. Je salue donc l'initiative du rapporteur Claude Kern de proposer comme nouvel intitulé : « Projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ». Cela nous semble plus fidèle au contenu, et je ne doute pas, madame la ministre, que vous partagerez ce point de vue. Pour la Pour la représentation nationale, l'examen de ce projet de loi est évidemment l'occasion d'évoquer la politique générale menée par le Gouvernement dans le domaine du sport. Dans cinq ans, en 2024, la France accueillera le monde, avec les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Le 13 septembre 2018, les sénateurs ont largement célébré cette attribution, en cohérence avec le soutien apporté depuis les prémices de la candidature de notre pays. Nous avons, par la suite, dès le premier semestre de 2019, adopté le projet de loi Olympique, d'adapter notre droit et de mettre en place un encadrement concret des procédures pour que nous puissions organiser dans les meilleures conditions le plus grand événement du monde, qui devrait attirer plus de deux millions de visiteurs et qui sera regardé par plus de quatre milliards de téléspectateurs dans le monde. Vous le savez, madame la ministre, le Sénat a une ligne de conduite : nous ne disons jamais oui par principe et jamais non par dogmatisme. Quand nous considérons qu'ils sont bons pour le pays, nous votons les textes ; dans le cas contraire, nous nous y opposons. Nous suivrons cette logique à propos du projet de loi que vous défendez aujourd'hui : je tiens d'ores et déjà à vous indiquer que le groupe Les Républicains n'y est pas opposé par principe. Nous considérons, cependant, qu'il est nécessaire

Cela étant dit, je souhaite vous faire part de notre vive inquiétude concernant l'avenir sportif de notre nation. La France est devenue une référence en termes d'organisation de grandes compétitions internationales, moment, le déroulement de la Coupe du monde de football féminin. J'en profite pour saluer le parcours de notre équipe de France, qui a suscité l'engouement des Français avant de chuter face au réalisme- certains de mes collègues diront peut-être l'impérialisme -américain. ans avant les Jeux de Paris, un an avant ceux de Tokyo, le Gouvernement ne cesse d'envoyer des signaux négatifs au milieu sportif. Ce projet de loi en est un nouveau. Je profite donc de ce débat pour appeler votre attention sur l'amendement que nous avons adopté jeudi dernier, sur l'initiative de notre collègue Michel Savin, qui, comme vous le savez, est particulièrement investi et réalise un formidable travail sur tous ces sujets. Un événement malheureux l'a contraint à ne pas être présent dans l'hémicycle aujourd'hui. Ce dispositif, introduit par le Sénat dans le projet de loi de transformation de la fonction publique, concerne les conseillers techniques sportifs. Vous vous étiez engagée, madame la ministre, à ne pas utiliser à leur égard le dispositif de détachement d'office auprès des fédérations. Nous avons donc souhaité traduire cet engagement dans la loi, mais l'avis défavorable du Gouvernement ne nous rassure pas sur ses intentions. Nous voulons bien vous croire sur parole, toutefois, pourquoi inscrire un tel dispositif dans le marbre de la loi si vous n'entendez pas l'utiliser ? Nous pourrons éventuellement discuter de nouveau de ce sujet dans un futur texte, par exemple lors de la grande loi sur le sport que l'on nous promet et que nous attendons ici impatiemment. il faut apaiser et donner des signes de bienveillance au mouvement sportif et à ses personnels, qui, au quotidien, préparent nos athlètes et participent au déploiement de la politique sportive dans nos territoires pour tous les publics. Le Sénat a, encore une fois, apporté la preuve de son soutien au mouvement sportif, et je pense qu'il serait incompréhensible que votre majorité revienne sur cette avancée. Je tiens aussi à rappeler le très gros investissement du Sénat en faveur de la politique sportive française, que, malheureusement, le Gouvernement ne soutient pas complètement. Sortons des positions dogmatiques pour que la France tienne son rang de grande nation sportive, comme le souhaite le Président de la République. Ainsi, le Sénat augmente chaque année le budget des sports et, chaque année, le Gouvernement le rejette. Je veux bien tout entendre, mais on ne peut pas décemment soutenir que ce budget a été « préservé », selon vos termes, alors qu'il accuse une baisse de 6 % par rapport au dernier exercice. Par ailleurs, le Sénat a adopté, dans le projet de loi pour une école de la confiance, des dispositifs ambitieux pour une pratique quotidienne des activités physiques et sportives à l'école ainsi que pour l'accompagnement des jeunes souhaitant accéder au plus haut niveau sportif. Las, la majorité gouvernementale n'en a soutenu aucun lors de la commission mixte paritaire. Enfin, il y a deux semaines, le Sénat a inscrit dans les missions de la future Agence nationale de la cohésion des territoires le soutien aux politiques de la culture et du sport, terreau indispensable à la cohésion sociale. Le Gouvernement soutiendra-t-il cette mesure ? S'agissant du projet de loi en discussion,

Cette dissimulation initiale souligne certainement la fébrilité du Gouvernement à ce sujet, et nous ne pouvons que le regretter. Cela cacherait-il d'autres intentions moins louables ? Comme un grand nombre de mes collègues, je m'interroge sur votre objectif à terme. En confiant à cette agence des missions qui relevaient jusqu'à présent du ministère des sports, ne risque-t-on pas de vider celui-ci de sa substance et,, de programmer sa disparition pure et simple ? Sans parler de privatisation rampante du service public- j'en laisserai le soin à d'autres -, je m'inquiète du transfert décisionnel vers des instances qui échapperont à un contrôle digne de ce nom. Le groupe Les Républicains du Sénat soutient le principe d'une évolution du modèle sportif qui a été mis en oeuvre par le général de Gaulle. Cependant, celui-ci a fait ses preuves, et il est envié par de nombreuses nations dans le monde ; si l'objet de ce texte est de réformer pour réformer, par pur principe, ce n'est pas une bonne chose. Le ministère des sports a son utilité, nous en sommes convaincus, comme nous sommes convaincus des bienfaits d'une gouvernance partagée et d'un pouvoir plus important confié aux fédérations, notamment concernant le haut niveau. Depuis janvier 2018, de nombreuses tables rondes et ateliers ont été organisés, ce qui a permis à l'ensemble des acteurs de discuter et de travailler à un nouveau modèle plus coopératif et à une gouvernance partagée entre l'État, le le mouvement sportif, le monde économique et les collectivités territoriales, dont je veux à mon tour rappeler qu'elles sont les véritables financeurs du sport en France, avec plus de 12 milliards d'euros annuels de dépenses. Ces différents acteurs ont réussi à aboutir à un accord de gouvernance partagée, au sein d'une agence qui aura la charge du haut niveau et de la pratique quotidienne pour tous. J'en profite pour rappeler, et ce n'est pas le moindre des griefs, qu'à aucun moment les parlementaires n'ont été associés à ces travaux. Nous votons pourtant le budget des politiques publiques sportives et nous en contrôlons l'utilisation ; nous sommes également quotidiennement au contact des acteurs de terrain du milieu sportif. Nous ne pouvons que regretter que, sur un sujet si important pour la France, la représentation nationale n'ait même pas été interrogée.

La structure existe donc, mais son fonctionnement demeure très flou, et personne n'est aujourd'hui en mesure de nous expliquer concrètement comment cette agence se déclinera sur les territoires, ni quelle sera la répartition exacte entre les missions qui lui seront attribuées et celles que vous conserverez.

Allez-vous suivre ses recommandations ? Alors que le modèle de l'agence est censé être un héritage des jeux de 2024 pour notre pays, circonscrire sa durée de vie remettrait en cause cet objectif et rendrait encore plus incompréhensible sa mise en oeuvre. oeuvre. Ensuite, avec votre majorité, allez-vous soutenir le dispositif adopté en commission pour permettre à des parlementaires de siéger au sein de l'agence ? Là aussi, nous entendons un double discours : alors que la proposition de loi déposée par notre collègue Michel Savin en février dernier a été largement soutenue sur nos travées,

Enfin, je voudrais insister sur la déclinaison territoriale de l'agence. En premier lieu, le délégué territorial de l'agence devrait être le préfet de région : pourquoi pas. Je tiens à apporter mon soutien à la circonscription de leur rôle adoptée en commission sur l'initiative de notre rapporteur. Néanmoins, cette mesure recentralise, en quelque sorte, le dispositif de l'agence, ce qui va à l'encontre de la gouvernance partagée mise en oeuvre au niveau national. Nous avons bien compris que le Gouvernement et l'État essaient par tous les moyens de remettre en question le réel partage de la gouvernance, mais il faut donner aux acteurs les garanties que celle-ci sera réellement partagée, tant au niveau national qu'au niveau territorial.

sportive, je ne saurais trop vous prier de prendre la balle au bond, car, pour faire référence à votre ancienne spécialité, je suis convaincu que vous n'avez nullement pour objectif de couler l'élite du sport français, ni de vous mettre à dos l'ensemble des acteurs du monde sportif

introduire la notion de stricte proportionnalité entre les mesures qui seront prises pour limiter la circulation la délimitation de voies réservées et les besoins réels de circulation des véhicules accrédités. Je rappelle que, outre

Ouzoulias, pour explication de vote.

vous nous demandez, par cette loi d'exception, d'organiser les pouvoirs spéciaux du préfet de police pour permettre la relégation des populations de Seine-Saint-Denis sur des voies annexes, afin de laisser le passage libre aux convois officiels. La proportionnalité,

pour déterminer la durée de mise en service des voies olympiques risque de favoriser les contentieux sur les dates de mise en service de ces voies, alors que l'ordonnance contient déjà une garantie très forte et très claire sur la durée de réservation des voies olympiques, laquelle ne sera possible que du 1juillet au 15 septembre. En outre, une distinction sera faite entre des voies

des membres de la famille olympique. Il nous paraît donc indispensable de ne pas modifier l'ordonnance sur ce point, afin d'assurer la sécurité juridique des voies olympiques.

consultation obligatoire est donc inutile. Je répète qu'il nous paraît indispensable de ne pas modifier l'ordonnance du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

qui seront utilisées pour la tenue des jeux Olympiques, il y a actuellement plusieurs détenteurs de l'autorité de police de la circulation et du stationnement. Il est prévu d'opérer une

Ce que la commission des lois vous demande, c'est simplement de ne pas oublier que, dans la gestion des espaces publics, les collectivités territoriales ont un petit rôle à jouer ... Le moment venu, vous serez

où il s'agit seulement, comme la rapporteur pour avis de la commission des lois l'a expliqué, d'assurer une parfaite collaboration entre les autorités compétentes ? Au reste, elle a rappelé que la procédure de consultation des autorités normalement détentrices du pouvoir de police de la circulation s'applique déjà, à Paris,

La rédaction de la commission est à nos yeux restrictive, car elle exclut

La Constitution séparant nettement les domaines de la loi et du règlement, procéder ainsi n'était pas possible. Nous avons donc introduit une nouvelle

Se limite-t-elle à l'organisation de déjeuners très médiatisés avec nos meilleurs sportifs et à la remise de Légions d'honneur à l'Élysée ? Je suis volontairement taquin et caricatural, mais, madame le ministre,

de reconnexion sociale. Nous l'avons tous constaté : alors que l'école est de moins en moins un lieu de mixité sociale, c'est encore le cas des clubs sportifs. Certes, le sport, les éducateurs, les extraordinaires bénévoles des clubs ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de notre société, mais ils offrent des bienfaits dont il serait dramatique de se passer. Ces clubs sportifs, ces stades sont d'extraordinaires lieux d'échanges et même de brassage social autour d'une même passion. C'est clair ! Combien de membres de la même association, issus cependant de milieux sociaux et culturels différents, ne se seraient peut-être jamais rencontrés sans le sport ? Quelques sages amendements permettront d'améliorer ce texte, mais c'est une vraie loi spécifique

Le Gouvernement ne les a pris que très partiellement en compte. Ainsi, la forme du GIP ne devrait concerner que des organismes chargés de mettre en oeuvre des projets temporaires, en aucun cas un organisme chargé d'appliquer des politiques publiques de façon permanente.

face à cette dérive : ne rentrez pas dans l'histoire du sport français comme la ministre du sabordage d'un système qui a permis votre parcours exceptionnel

vaudra pour demain, sans doute pour après-demain, mais certainement pas après les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : une fois la flamme olympique éteinte, on parlera vite de feu le ministère des sports

Je peux vous dire, madame la ministre, que le monde sportif est inquiet pour l'avenir. Sans s'accrocher au passé, force est de constater que notre modèle sportif, certes perfectible, a produit dans le passé des bienfaits. La réforme proposée tend à rompre avec une organisation du sport de haut niveau et du sport de masse qui date, dois-je le rappeler, de Léo Lagrange, le flambeau ayant ensuite été repris par Maurice Herzog, Alain Calmat, Marie-George Buffet et, plus récemment, Patrick Kanner. Enfin, je note une contradiction entre, d'une part, les ambitions louables affichées par le Président de la République et par le Gouvernement en termes de résultats et de médailles,

J'ai lu avec attention l'étude d'impact qui accompagne ce projet de loi : à la page 9, il y est écrit que, « de fait, tous les pays qui ont confié la mission d'améliorer les performances de leurs athlètes à une organisation autonome [ ...] ont vu leur performance aux jeux Olympiques et Paralympiques augmenter significativement. À

Le scrutin est ouvert.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

d'appliquer un principe de précaution pour que soient prises en compte toutes les dimensions des activités physiques et corporelles. On pourrait débattre à perte de vue sur

? Cet amendement prévoit que l'ANS pourra également soutenir les projets développés par des acteurs privés. Cette possibilité n'est pas exclue par la rédaction de la commission, qui comporte

Lozach. Cet amendement vise à permettre à l'ANS de collecter tout type de ressources auprès de personnes morales, tant de droit public que de droit privé. Il s'agit tout simplement d'élargir les sources de financement de l'ANS afin qu'elle puisse collecter des recettes de mécénat ou de sponsoring et bénéficier de subventions, de dons ou de legs.

Monsieur le sénateur, vous souhaitez que, au-delà des ressources classiques actuellement prévues par la loi pour un GIP, l'agence puisse bénéficier d'un panel de ressources élargies. Il est à notre avis tout à fait souhaitable que l'ANS puisse diversifier ses sources de financement.

Il est proposé d'en faire l'ordonnateur des dépenses et le responsable de la mise en oeuvre de concours financiers territoriaux de l'agence. Ces précisions sont utiles. les missions de l'ANS ne se limitant pas exclusivement au développement du sport pour tous dans les territoires les moins favorisés, il ne convient pas d'inscrire cette précision dans la loi.

Faute de précision, les craintes relatives à une recentralisation rampante ne pourraient que perdurer, et la confiance en l'ANS se trouverait dès lors fragilisée. Plus globalement, cela rejoint la préoccupation de la commission de faire figurer dans la loi les garanties nécessaires concernant la gouvernance territoriale de l'agence. La suite de la navette devra permettre de préciser la rédaction de l'article 3 sur ce sujet. Dans cette attente, j'émets, à titre personnel,

Avis favorable également

proposons de préciser qu'elle devra agir en coordination avec les instances de direction de l'ANS. Ces conférences régionales seront en quelque sorte des émanations de l'Agence nationale du sport,

Mireille Jouve. La rédaction initiale du projet de loi était silencieuse sur la place allouée aux collectivités territoriales au sein de la future Agence nationale du sport. Nous saluons une nouvelle fois la volonté du rapporteur de favoriser un débat parlementaire sur l'ANS. Acteurs majeurs du sport, les collectivités territoriales

et d'être les lieux d'élaboration des nouvelles politiques de réduction des inégalités ou des nouvelles pratiques territoriales à développer. À cette fin, il convient que leur présidence soit assurée par un représentant des collectivités territoriales, des EPCI

Il semble préférable de ne pas exclure la possibilité qu'un représentant du mouvement sportif puisse également être désigné, comme le prévoit l'amendement n° 16 rectifié. L'essentiel est que ces instances ne soient pas animées par des représentants de l'État, dont le rôle est différent. La commission

Même si le texte de la commission ne le prévoyait pas explicitement, c'est tout à fait dans l'esprit de sa rédaction. L'avis est donc favorable.

Mme Mireille Jouve. En matière de représentativité, les associations départementales de maires ou de présidents d'EPCI sont des outils précieux sur lesquels nous pouvons, une nouvelle fois, nous appuyer. Elles sont un relais fidèle des doléances des communes et des intercommunalités.

les représentants des collectivités locales soient désignés par la ou les associations départementales de maires et de présidents d'intercommunalité les plus représentatives. Le dispositif de l'amendement présenté par Mme Jouve

aux associations représentatives, alors que la rédaction adoptée par la commission renvoie, par souci de souplesse, à un décret en Conseil d'État. Faut-il inscrire dans la loi le rôle des associations représentatives ? Je pense que les modalités de fonctionnement de la gouvernance territoriale de l'ANS feront encore l'objet de discussions entre les acteurs. Néanmoins, pour des raisons pratiques, il est évident que les associations d'élus auront un rôle à jouer dans la désignation des représentants des élus au sein de la conférence régionale du sport. La commission émet un avis favorable

l'avis de la commission ? L'organisation des conférences des financeurs au niveau territorial est un sujet complexe, qui fait l'objet d'une concertation. Autant il semble utile d'en fixer les principes essentiels dans la loi, autant il apparaît prématuré de prévoir prévoir dans celle-ci un mécanisme de repli au niveau départemental en cas d'échec au niveau local. Par ailleurs, la comparaison avec les CTAP ne semble pas

Au vu de la nature d'une convention d'objectifs dont la durée est par ailleurs déjà fixée, il ne semble pas nécessaire de prévoir dans la loi son contenu et son cadre pluriannuel. En outre, l'agence occupera déjà une place importante dans les documents budgétaires soumis au Parlement

Ce n'est évidemment pas la même chose ! La rédaction adoptée par la commission s'inspire des contrats d'objectifs et de moyens existant entre l'État et les sociétés de l'audiovisuel public. Le processus est connu ; il permet en particulier de définir des moyens de manière pluriannuelle. On ne peut que s'inquiéter du refus du Gouvernement de s'engager sur des objectifs pluriannuels de financement de l'agence. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'avenir du sport et cela renforce les inquiétudes liées au manque de moyens de l'agence à son lancement. La navette permettra, je l'espère, d'améliorer la rédaction de cette disposition. Pourquoi, par exemple, vouloir supprimer la présentation du rapport annuel devant les commissions ? En l'état actuel des choses, il me semble préférable de maintenir la rédaction de la commission. C'est pourquoi, à titre personnel, je suis défavorable

est à M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le conseil d'administration de l'agence comprendra deux députés et deux sénateurs nommés par les présidents de chacune des assemblées. Compte tenu des dispositions de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018, il n'apparaît pas nécessaire de mentionner le respect de la parité ou du pluralisme dans les nominations, dans la mesure où il s'agit déjà d'obligations légales.

présence apparaît d'autant plus justifiée que les entreprises sont des acteurs importants du financement du sport, à travers les droits télévisés, les partenariats et la publicité.

Personnellement, je comprendrais très mal qu'une structure dans laquelle on trouve des représentants du monde économique, parmi lesquels le Medef, la Confédération des PME ou l'Union Sport et Cycle,

Le milieu des CTS est très disparate et hétérogène ; il comprend notamment des conseillers d'animation sportive, qui sont en phase directe avec les clubs et ne sont pas véritablement impliqués dans la préparation olympique.

dispositif confiant au responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport la compétence pour l'affectation des CTS, leur formation et leur évaluation, dispositif qui vient modifier le statut des CTS

qu'il est d'accord pour préserver l'alinéa 11 de l'article 28 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture ? Dans ce cas, nous pourrions renoncer à l'alinéa 41

Dans ces conditions, il est selon moi indispensable de prévoir, à titre de précaution, que c'est le responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport qui aura pour mission d'affecter les CTS aux fédérations, ce qui constituera un verrou face au projet de transfert obligatoire des CTS.

garder la main sur le service public du sport au travers des CTS, qui sont votre bras armé pour mener à bien les politiques décidées par l'État. Nous entendons graver dans

pour qualifier les besoins et apporter des réponses sur mesure et réactives aux acteurs de la performance » et « en complément ou en remédiation lorsque les conditions de préparation ne permettent pas de tenir la promesse de performance et de résultats Compte tenu de cette implication opérationnelle dans la recherche de la performance sportive, le présent amendement vise à étendre aux organes et aux préposés de l'Agence nationale du sport des obligations pèsent actuellement sur ceux des fédérations sportives en matière de signalement de faits de dopage à l'Agence française de lutte contre le dopage et de coopération aux enquêtes menées par celle-ci.

Les titulaires de ces contrats sont sélectionnés à l'issue d'une procédure organisée par le COJO et présentant toutes les garanties d'impartialité, de transparence et de publicité. Il serait donc redondant de demander au COJO de respecter une seconde fois, lorsqu'il accordera des titres de sous-occupation du domaine public à ses partenaires, des exigences déjà satisfaites au moment de leur sélection. La loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a explicitement exclu de l'application des règles de la commande publique la délivrance de titres de sous-occupation du domaine public aux partenaires désignés par le Comité international olympique. Il convient de faire de même pour les partenaires du COJO. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement l'avis de la commission ? Cet amendement vise à modifier les dispositions de l'article 17 de la loi du 26 mars 2018, relatif aux règles applicables au COJO en matière de marchés publics.

Michel Laugier, pour explication de vote.

loi. M. Robert Navarro a fait connaître à la présidence qu'il se démettait de son mandat de sénateur de l'Hérault à compter du 30 juin 2019, à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il est remplacé par Mme Agnès Constant, dont le mandat de sénatrice a commencé le 1 juillet 2019, à M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 1 juillet 2019 et complétant le décret du 17 juin dernier portant convocation du Parlement en session extraordinaire. Acte est donné de cette communication. Ce décret a été publié sur le site internet du Sénat. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte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

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires (proposition n° 168, texte

Rousseau rassemblait sous le vocable d'éducation « tout ce que nous n'avons pas à notre naissance et dont nous avons besoin étant grands ». L'éducation est le lieu où se structure l'identité du jeune enfant, où s'affirment son libre arbitre et sa capacité de jugement. En cela, le temps éducatif est vécu, tant du côté de l'enfant que de celui de l'adulte, comme un apprentissage où chacun s'expose à l'autre et confronte ses représentations, ses désirs. Dans la relation éducative, le parent doit savoir se faire pédagogue. On ne peut élever un enfant sans se référer à des principes, à des savoir-être. L'objectif est immense : faire de l'enfant un être autonome, capable de socialité, portant au coeur l'idéal de fraternité. La qualité première du pédagogue, c'est d'avoir le souci constant de la cohérence entre les principes affichés et les méthodes employées. L'ascendant de l'adulte sur l'enfant est, dans ces circonstances, inévitable. Il a le devoir de fixer le cadre éducatif. Tout le paradoxe est là : l'autonomie de tout enfant se construit dans la dépendance.

Le parent accompli, comme le bon éducateur, doit savoir faire oublier la tutelle qu'il exerce sur son enfant. Les violences éducatives, à l'inverse, exacerbent cette relation d'assujettissement : elles ont souvent des effets irréversibles chez l'enfant ; elles sont souvent le symptôme symptôme des difficultés rencontrées par les parents dans l'éducation de leurs enfants. « Il y a beaucoup de choses terribles dans ce monde, mais la pire est qu'un enfant ait peur de son père, de sa mère ou de son professeur a écrit Janusz Korczak, l'un des plus grands pédagogues du siècle dernier. Agnès Buzyn l'a rappelé au mois de novembre dernier : on n'éduque pas par la peur. La peur, on s'y enferme et on y étouffe. Les coups, les raclées, les fessées sont autant de stigmates que l'enfant devra porter toute sa vie. Je rappellerai ces chiffres, terribles, qui nous permettent de prendre la mesure de l'ampleur du phénomène selon la Fondation pour l'enfance, 85 % des parents français ont déjà eu recours à des violences éducatives ordinaires ; 75 % des maltraitances infantiles sont le fait de « punitions éducatives corporelles ; plus de 50 % des parents ont frappé leur enfant avant l'âge de deux ans, persuadés que l'éducation qu'ils avaient eux-mêmes reçue leur avait été utile et profitable. Rien n'est plus faux que l'idée selon laquelle les violences éducatives ordinaires « forgeraient le caractère

nous savons aujourd'hui qu'une éducation punitive a des conséquences désastreuses sur le développement, la santé mentale et la stabilité affective de l'enfant. Des conséquences à la fois immédiates et de long terme sont observées : elles portent sur toute la vie du sujet qui aura eu à essuyer des humiliations et des châtiments corporels dans sa prime enfance. À court terme, on observe une hausse des comportements agressifs chez les enfants ayant subi des violences, un risque accru de troubles cognitifs. À long terme, on peut observer une baisse de l'estime de soi, des comportements antisociaux, une augmentation de la prévalence de troubles mentaux et addictifs et, pour les cas les plus graves, une déficience mentale liée à une réduction de la zone grise du cerveau, un risque d'obésité plus élevé ainsi que des troubles cardiovasculaires. Les anciens enfants battus,

auxquels ils se sont trouvés exposés. Les enfants victimes de violences familiales sont susceptibles de devenir des adultes constamment habités par la peur et l'insécurité.

Il y a urgence à agir et à voter une proposition de loi d'interdiction des violences éducatives ordinaires. Ce vote permettra à notre pays de faire un pas de plus vers la traduction effective de ses engagements internationaux dans le droit interne. Il y a, dans notre pays, une absence d'interdiction formelle des violences éducatives ordinaires en droit interne, où subsiste encore dans la jurisprudence un « droit de correction » totalement anachronique.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

le droit des parents à faire souffrir leurs enfants. Notre rôle est d'exiger, au nom des enfants, de leur intérêt supérieur, un droit absolu à la dignité et à l'intégrité physique. C'est là un signal, que certains jugeront symbolique, mais en réalité extrêmement fort, adressé aux jeunes et futurs parents de notre pays. Ce que nous souhaitons, c'est promouvoir une éducation bienveillante, fondée sur la confiance, le dialogue et le respect mutuel. Janusz Korczak aimait à comparer l'enfant à cet étranger plongé « dans une ville inconnue dont il ne connaît ni la langue, ni les coutumes, ni la direction des rues Pour s'orienter, l'enfant a besoin de repères, il doit pouvoir trouver une oreille attentive et une main réconfortante tout au long de sa vie, une vie faite de joies et d'erreurs, car l'erreur est le sel de l'apprentissage. Nos maîtres d'école ressassaient que la répétition est l'art de la pédagogie. Cet art requiert de la patience, de la méthode, une attention quasiment éthique portée à l'autre : en un mot, de l'amour. C'est d'ailleurs ce terme qu'emploie le préambule de la Convention internationale des droits de l'enfant pour décrire l'atmosphère familiale dans laquelle devrait grandir chacun de nos enfants.

C'est le sens de la politique de « soutien à la parentalité » que je mène à la tête du secrétariat d'État à la protection de l'enfance. Je partage, avec mes collègues du ministère des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn et Christelle Dubos, cette conviction simple : on ne naît pas parent, on le devient. L'apprentissage de la parentalité relève d'un équilibre subtil entre confiance en soi et capacité à répondre aux besoins de l'enfant. Les violences éducatives sont l'expression d'un déséquilibre affectant la nature même de la relation entre les parents et leurs enfants. La prévention des difficultés éducatives des parents constitue le socle de la politique de protection de l'enfance. Je veux croire qu'une politique de soutien à la parentalité efficace rendrait superflues- dans un monde idéal, peut-être -les mesures de protection.

Cet accompagnement, c'est le coeur du volet préventif de notre politique de l'enfance : protéger les enfants, cela commence parfois par mieux accompagner les parents dans leur projet d'être parents. C'est tout l'objet

c'est sans doute lors de ces 1 000 premiers jours que le parent a le rôle le plus décisif et que pèsent parfois sur lui les plus grandes appréhensions : comment donner la première tétée, puis le premier biberon ? Que faire face à un bébé qui ne cesse de pleurer ? Pourquoi ne faut-il pas le secouer ? Comment faire concorder le cycle de vie du bébé avec ses propres impératifs ? Pourquoi ne pas l'exposer aux écrans ? Pourquoi lui offrir une éducation bienveillante ? Notre mission d'accompagnement est à ce titre essentielle, voire vitale en ce qui concerne la prévention du syndrome du bébé secoué. Je conçois cette politique de soutien à la parentalité comme reposant sur deux outils majeurs d'une part, une protection maternelle et infantile mieux soutenue financièrement et rebâtie autour de ses missions historiques de prévention- je pense notamment aux visites à domicile maternelles et préventives ou à la mise en place d'un entretien prénatal obligatoire au quatrième mois de grossesse,

Le vote de cette proposition de loi constituera, à ce titre, une avancée importante. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a aussi vocation à graver dans le marbre

Être parent, c'est être garant du respect des droits de ceux qui sont à sa charge. Être parent, c'est respecter l'enfant pour ce qu'il est, et aussi en tant qu'être en devenir. L'enfance est un âge de la vie, avec ses valeurs, ses sensibilités, ses aspirations et ses stratégies sociales. L'enfant n'est en aucun cas inférieur à l'adulte : une telle conception de l'enfance

la sanction étant plus élevée encore s'agissant d'une victime mineure de 15 ans ou moins. Le message de prohibition figurera, grâce à l'adoption de cette proposition de loi, dans le code pénal, en appui de l'article 222-13. Pour lui donner une meilleure visibilité, nous le ferons également figurer en première page des carnets de santé. Le poids de la culture et des traditions n'est pas négligeable. La violence est alimentée, confortée par une certaine tolérance de l'opinion publique.

de changer les pratiques et le regard de nos concitoyens sur les faits de maltraitance. Nous devons désormais parler d'aventure éducative. On peut, à ce titre, se remémorer les très belles lignes de Janusz Korczak pour entrevoir le plus beau et difficile métier de parent de parent : « Vous dites : c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez : parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt le fait d'être obligé de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. messieurs les sénateurs, j'aimerais vous dire la fierté qui est la mienne d'être devant vous aujourd'hui pour soutenir, au nom du Gouvernement, cette proposition de loi. Elle répond à notre engagement en faveur d'une société sans violences faites aux enfants, d'une société plus attentive à la place et à la parole de l'enfant.

-et l'affirmation de la non-violence comme principe d'éducation. Ces textes répondent à une attente et à une évolution nécessaire de la société. Ils s'inscrivent aussi dans la continuité de deux lois importantes en matière de protection de l'enfance : celle du 5 mars 2007, portée par notre président de la commission des lois, Philippe Bas-

Chacun sait que la violence ne peut être un mode d'éducation. Pourtant, ces violences que l'on qualifie d'« éducatives » et d'« ordinaires » sont encore aujourd'hui communément admises, voire justifiées. Il est en effet établi que 85 % des parents y ont recours dans l'éducation de leur enfant, et dans plus de 50 % des cas avant l'âge de 2 ans. Ces chiffres montrent combien ces pratiques sont encore largement répandues. Nous ne devons pas les minimiser, même si, bien sûr, et c'est heureux, les mentalités évoluent progressivement. Ils montrent, aussi et surtout, combien une prise de conscience collective est nécessaire. se fait peu à peu, repose sur l'affirmation d'un principe simple : la violence n'est pas acceptable, qu'elle soit exercée envers un adulte ou envers un enfant. C'est tout le sens de la démarche législative qui a été entreprise conjointement par l'Assemblée nationale et le Sénat. Depuis près de vingt ans, les recherches scientifiques ont mis en évidence les conséquences néfastes de ces violences pour l'enfant. Des travaux en neurobiologie ont démontré que l'exposition au stress fragilise le développement cérébral de l'enfant, ce qui peut favoriser des troubles de l'apprentissage ou de la mémorisation, et que les violences peuvent conduire l'enfant à intérioriser l'idée d'une violence admise, tolérée à l'encontre des personnes proches, susceptible de constituer un mode de résolution des conflits.

à modifier et à compléter l'article 371-1 du code civil. Elle comporte également deux articles, de portée plus secondaire, sur lesquels je reviendrai. Rappelons que l'article 371-1 du code civil

permettra d'accompagner le changement social déjà à l'oeuvre et de lui donner un fondement juridique. Inscrire dans la loi de façon explicite l'interdiction de toute violence permettra aussi une évolution de la jurisprudence que j'évoquais, qui ne pourra qui ne pourra plus s'abriter derrière un attribut implicite de l'autorité parentale pour justifier l'existence d'un « droit de correction ». Poser le principe de cette interdiction permettra

énoncée spécifiquement dans la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a ratifiée en 1990 et dont on fête cette année le trentième anniversaire. Cette convention prévoit une obligation, pour les États parties, de prendre toutes mesures législatives « pour protéger l'enfant contre toute forme de violence,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

assemblée est peu disposée à voter des demandes de rapport, mais, le président Bas nous le rappelle souvent, le Gouvernement n'étant pas dans l'obligation constitutionnelle

la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise vise à inscrire dans le code civil le principe selon lequel l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Cette proposition de loi prévoit la formation des assistantes maternelles à la prévention des violences éducatives ordinaires. Elle comporte aussi une demande d'un rapport dressant un état des lieux des violences éducatives

Au mois de mars dernier, déjà, nous avions examiné et adopté un texte similaire, déposé par notre collègue Laurence Rossignol. Aujourd'hui, nous sommes saisis d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par la députée Maud Petit.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

cette proposition de loi suscite au sein du groupe Les Indépendants un sentiment très mitigé. Toutefois, il apparaît inutile de prolonger la navette sur un texte dont la disposition centrale, à l'article 1, a déjà été adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées. de loi s'inscrivant dans le prolongement des lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 relatives à la protection de l'enfance, son adoption sans délai mettra la France en phase avec la majorité de ses partenaires européens.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour débattre de l'interdiction des violences éducatives ordinaires, quatre mois seulement après avoir voté une proposition de loi socialiste quasiment identique Aussi, mes chers collègues, je m'interroge : que doivent penser nos concitoyens du temps que nous passons à ressasser les mêmes questions ? Ne devrions-nous pas consacrer notre précieux temps législatif à d'autres sujets qui préoccupent réellement les Français ?

Une nouvelle fois, on s'amuse avec le sujet de la fessée, mais on ne propose rien de concret pour empêcher et sanctionner la vraie violence. Notre position est la même qu'il y a quatre mois : cette proposition de loi n'apporte rien de révolutionnaire.

notre droit permet déjà de sanctionner et de condamner les parents qui se rendraient coupables de maltraitance. Est-il nécessaire d'en rajouter ? Je n'en suis pas certaine ... Il suffit d'appliquer

N'est-ce pas là la fonction d'un discours politique plutôt que d'un article du code civil ? La loi ne doit pas être seulement symbolique, elle doit avoir une portée certaine. Le dispositif proposé soulève une autre difficulté : que sont précisément les violences éducatives ordinaires Veillons à ne pas confondre ce qui relève de la maltraitance avec ce qui vise à mettre un terme à certaines pratiques des enfants. À un moment donné, il faut bien leur dire « non ». N'est-ce pas un certain François Bayrou, alors candidat à l'élection présidentielle, qui, en 2002, avait giflé un enfant dans la rue pour l'empêcher de lui faire les poches ? Doit-on bannir toute éducation qui pourrait comporter parfois, sans forcément une intention évidente des parents, un geste ferme pour indiquer à un enfant de ne pas toucher aux plaques de cuisson chaudes, aux produits ménagers ou aux prises électriques ? Quels gestes relèvent des violences ? Quels gestes sont au contraire « tolérables » ? La rédaction proposée est peu intelligible de ce point de vue. Une fois de plus, son application, alors qu'elle a vocation à clarifier une jurisprudence, ne semble pas évidente. Si le droit n'est pas clair, comment espérer son application uniforme ? Enfin, les Français en ont assez de cette ingérence de l'État, qui voudrait les « rééduquer » et leur dire comment éduquer leurs enfants. L'éducation relève en premier lieu des parents et du cercle familial. Être mère, être père, c'est une responsabilité. Elle doit être assumée pleinement.

J'espère toutefois qu'il ne restera pas lettre morte et que son adoption aboutira à la mise en place de dispositifs concrets de soutien à la parentalité. Mes chers collègues, je pense qu'il est temps de cesser d'opposer les « bons », qui seraient contre les violences, et les « méchants », qui seraient pour. Nous sommes tous opposés aux « vraies » violences contre les enfants. Nous sommes tous favorables aux initiatives qui visent à préserver le bien-être de l'enfant et son intérêt. Nous sommes tous convaincus que l'éducation est un sujet crucial, au fondement même de la société. Par souci de cohérence, nous voterons ce texte, car il correspond peu ou prou à ce que nous avons voté voilà quatre mois. Même s'il revêt un caractère essentiellement symbolique, il a au moins le mérite de rappeler une règle de bon sens, dont la violation est déjà sanctionnée par la loi. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, pour la seconde fois en l'espace de quelques mois, notre assemblée examine un texte dont l'objet est de faire reculer les violences éducatives en inscrivant dans notre droit civil le principe d'une autorité

Notre groupe approuve pleinement cette modification du code civil. Elle est bien plus que symbolique, puisque le juge pénal, le juge aux affaires familiales et le juge des enfants pourront s'appuyer sur cette définition utilement complétée de l'autorité parentale.

des violences éducatives sur le développement de l'enfant : atteinte à la confiance en soi, culpabilisation, troubles du comportement et de l'apprentissage, encouragement à percevoir la violence comme un mode acceptable de règlement des différends, potentielle transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Aussi est-il important d'être plus volontaristes encore pour informer et sensibiliser l'ensemble de notre société aux vertus d'une éducation bienveillante et non violente, ce qui n'exclut pas pour autant la discipline.

des assistantes maternelles en matière d'éducation sans violence, l'autre la remise d'un rapport par le Gouvernement. Notre groupe votera ce texte, en félicitant celles et ceux qui ont oeuvré au rapprochement des deux propositions de loi, au premier rang desquels Mme la rapporteure. La parole

Il est grand temps que la France se dote d'un dispositif législatif similaire et effectif. Tel est l'avis de nombreux neurologues et pédopsychiatres, selon qui l'interdiction des châtiments corporels et moraux

L'agressivité et les sévices habituent les enfants aux relations de domination et aux humiliations. Cette brutalité se répercute ainsi sur les rapports sociaux et s'étend à toutes les autres sphères de la vie sociale. Françoise Dolto, célèbre psychanalyste, déconstruisait déjà, au début des années soixante-dix, l'idée que l'éducation devait se conjuguer avec l'autorité et la punition. Ses travaux ont permis à l'enfant d'accéder au statut de personne à part entière. Trente ans après son décès, nous sommes enfin prêts à inscrire dans la loi l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Longtemps, nous avons toléré le « droit de correction » dans la sphère familiale et dans les milieux éducatifs. Cette acceptation, consciente ou inconsciente, relève des derniers vestiges du patriarcat et d'une époque où où la soumission au était culturellement la règle. Ce « droit de correction », admis par la jurisprudence, nous a valu de nombreuses condamnations par les instances européennes pour non-respect des obligations en matière de protection des enfants. L'aide à l'enfance et la défense du mineur ne se limitent d'ailleurs pas à la sphère familiale. Que dire des mineurs étrangers isolés, des enfants placés et des pupilles de la Nation, qui subissent parfois de plein fouet une violence institutionnelle, doublée des violences éducatives ordinaires qui ont cours dans certains services de la protection de l'enfance ? Mes chers collègues, je souhaite vous rappeler les chiffres suivants : deux enfants meurent chaque semaine

tous les mineurs et ne se limite pas à la sphère familiale. Beaucoup reste encore à faire en la matière. Développons les services d'aide à la parentalité, et ce dans tous les milieux, aisés comme défavorisés. Quartiers huppés ou banlieues paupérisées, tous les territoires sont concernés. À celles et ceux qui objecteront que cette loi culpabilisera les parents, qu'il y a ingérence de l'État dans les relations intrafamiliales, je réponds par Il y a quelques décennies, on considérait aussi les violences faites aux femmes comme une affaire privée, un droit de correction marital. correction marital. Contrairement aux femmes qui, face à la violence conjugale, ont désormais la possibilité, même si cela n'est jamais aisé, de dire « non » et de menacer de partir ou de divorcer,

Si ce texte, accompagné d'une campagne de sensibilisation, peut permettre de faire évoluer les mentalités et de clarifier le rapport d'autorité liant les parents à leurs enfants, nous ne pouvons que le soutenir. La parole est à Mme Maryse Carrère.

il convient de l'écouter avec sérieux. Il est à égalité d'être avec un adulte, à ce titre il est un analysant à part entière. » Il faudra ensuite Il faudra ensuite attendre 1989 pour que soit adoptée la Convention internationale des droits de l'enfant, consacrant l'enfant comme une personne à part entière.

Cette prise en compte est primordiale, car elle intervient à une période essentielle de la construction de l'individu. C'est là qu'il acquiert des valeurs et des normes qu'il internalise et qui conditionneront l'adulte de demain. Depuis plusieurs années, les études le prouvent : le recours à la violence, notamment la fessée considérée encore comme une méthode éducative, favorise pourtant l'agressivité des enfants, conforte la baisse de leur estime et peut pénaliser leurs résultats scolaires. Plus alarmant, cette violence est parfois la porte d'entrée de châtiments plus graves. Aussi, il est important que nos enfants n'identifient plus la violence comme un mode d'éducation. Si certains pays comme la Suède ont légiféré à ce sujet depuis près de quarante ans, la France, elle, continue de violer ses engagements internationaux. Doit-on s'accommoder de cette loi du plus fort, où il suffit d'en venir aux mains pour régler un conflit et éduquer un enfant ? Si le code pénal interdit déjà toute forme de violence physique envers les enfants, notamment les plus jeunes, en en faisant une circonstance aggravante, rien n'est prévu à ce sujet dans le code civil. Cette proposition de loi, en prévoyant à l'article 371-1 du code civil que « l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques », vient clarifier la situation et poser un principe clair. Aucune éducation ne peut se faire par le châtiment corporel. En faisant un pas dans cette voie, la France honore enfin ses engagements internationaux. Ici, il s'agit de poser l'interdit de manière civile. Le but n'est pas de stigmatiser, ni de culpabiliser les parents, mais d'orienter vers un changement des pratiques sur le long terme. Le but n'est pas, comme nous avons pu l'entendre, de s'immiscer dans la vie familiale, mais bien de poser un interdit pour faire évoluer les mentalités dans un pays où 85 % des parents ont encore recours à la fessée. J'en conviens, l'éducation n'est pas toujours chose aisée, à une époque où les parents sont le plus souvent sous pression. Le lien familial s'est transformé ces dernières années, mais il est aujourd'hui nécessaire de faire évoluer de faire évoluer les modes d'éducation. De nombreux exemples montrent qu'il existe des méthodes plus douces et vertueuses pour se faire écouter des enfants. Si j'en reviens au texte, outre la disposition prévoyant que l'autorité parentale s'exerce sans violence, ce dernier prévoit également une sensibilisation aux violences éducatives ordinaires lors de la formation des assistants maternels. Ils peuvent ainsi mieux identifier l'impact de telles pratiques sur l'enfant et développer un environnement éducatif plus sain. Ce texte vient apporter de nouveaux droits aux enfants et prendre en compte leur intérêt supérieur, conformément à la convention internationale des droits de l'enfant. Comme l'avait dit ma collègue Josiane Costes lors de la lecture du texte proposé par notre collègue Laurence Rossignol, c'est aux magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation de se saisir de cette loi pour mettre fin à cette pratique d'un autre temps. Ma conviction profonde, c'est qu'il nous faudra à l'avenir être toujours plus vigilants sur les droits de l'enfant. Le récent rapport du Défenseur des droits sur ces sujets va d'ailleurs dans ce sens, en préconisant par exemple que les conseils départementaux ou les établissements hospitaliers désignent des référents en protection de l'enfance, ou en suggérant d'inscrire dans la loi l'interdiction de toute rétention administrative pour les familles avec enfants, Enfin, je rappellerai que notre intervention dans le domaine des droits de l'enfant est essentielle. Comme l'explique Pierre Verdier, nous sommes passés d'une conception d'intérêt de l'enfant à une définition des droits de l'enfant. Le droit, justement, vient alors comme un régulateur de pratiques. Il accompagne avant de sanctionner, il protège avant de punir et offre un cadre législatif pour une meilleure éducation. Je conclurai mon intervention par une remarque de forme : je trouve regrettable, en matière de travail législatif, que nous ayons eu à nous prononcer deux fois sur un texte quasi identique. Même si le temps législatif est long, j'espère qu'à l'avenir les différents groupes à l'Assemblée nationale comme au Sénat travailleront de concert afin que cette situation se reproduise le moins possible. Hormis cette remarque, vous l'aurez compris, l'ensemble des membres du groupe du RDSE approuvera ce texte qui marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance des droits de l'enfant. La parole

Face à un sujet sociétal aussi important que les violences éducatives ordinaires, il est regrettable d'assister à l'examen en parallèle de deux textes sensiblement identiques. Ce double débat est incompréhensible pour nos concitoyens c'est une perte de temps et cela abîme le Parlement. Quelle image renvoyons-nous quand, en mars dernier, nous avons examiné puis adopté- forcément -la proposition de loi de Mme Rossignol, alors que nous aurions pu adopter définitivement le texte de la députée Maud Petit Le Sénat et l'Assemblée nationale auraient pu sortir grandis, cela vient d'être dit, en démontrant leur capacité à s'unir sur ce sujet essentiel. Certes, monsieur le secrétaire

Aujourd'hui, il est donc temps de mettre fin à un débat qui a secoué sporadiquement notre pays pendant plusieurs décennies, débat qui s'est bien souvent résumé à des discussions de comptoir sur le thème « pour ou contre la fessée ? », tendant à rendre invisibles les autres violences, notamment psychologiques. Comme nous le rappelle la Fondation pour l'enfance, « violenter son enfant, c'est le marquer pour longtemps ». Aucun acte de violence n'est anodin. Aujourd'hui, l'idée a fait son chemin. Les parents aspirent à une nouvelle forme de parentalité, positive, et à une relation avec l'enfant construite sur la confiance et l'apprentissage. Nombre de livres, d'émissions, de podcasts traitent de la parentalité bienveillante. Une prise de conscience s'affirme : la violence n'est pas une pratique éducative. Parce que l'éducation joue un rôle fondamental non seulement dans la formation de l'être humain, mais aussi dans l'évolution de la société, il est primordial de l'exercer avec bienveillance.

Depuis quelques années, les neurosciences ont démontré les conséquences irréversibles de la violence sur les fonctions cognitives de l'enfant. On le sait, la maltraitance émotionnelle entraîne chez l'enfant un stress nocif pour le bon développement de son cerveau. Ce stress peut détruire des neurones qui jouent un rôle dans la mémoire, la gestion des émotions, la résilience et les capacités relationnelles. Par ailleurs, les neurones miroirs, l'enfant imite les parents.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 Un travail de sensibilisation de large envergure auprès des jeunes, futurs adultes et parfois futurs parents, reste également à imaginer, même s'il existe déjà des groupes de parole, des ateliers, des consultations aux centres

Enfin, cette semaine est importante pour la protection de l'enfance : après l'assemblée plénière du Conseil national de la protection de l'enfance, hier, l'adoption définitive de cette proposition de loi, aujourd'hui, les Assises nationales de la protection de l'enfance auront lieu les 4 et 5 juillet prochains à Marseille. Des annonces sont attendues

Cette proposition de loi s'inscrit dans l'histoire. Nous rejoindrons ainsi les cinquante-quatre pays dans le monde qui se sont déjà dotés d'une telle loi, quarante ans après la Suède qui en ouvrait la voie. Le groupe Union Centriste votera en faveur de cette proposition de loi.

L'opinion publique est régulièrement choquée par le décès d'un enfant sous les coups de ses parents. Si, heureusement, les violences intrafamiliales ne tuent pas toujours, les spécialistes sont unanimes quant aux dégâts qu'elles occasionnent sur les enfants qui en sont les victimes. Pour appeler l'attention de tous sur cet enjeu considérable, il faut compléter la définition de l'autorité parentale prévue à l'article 371-1 du code civil en précisant que,

et à la citoyenneté visant à interdire la pratique des violences dites « éducatives ordinaires ». Nous avions souligné alors l'immense portée symbolique de cet article du code civil. Lu dans toutes nos mairies à l'occasion des mariages, il est entendu par toute l'assistance, forcément attentive, attentive, en ces moments solennels, à la manière dont les familles se créent. Cette avancée ne fut qu'une victoire de courte durée. Le Conseil constitutionnel, saisi par certains d'entre vous, a censuré cette disposition, préférant conserver, dans l'intimité de chaque famille,

Au Sénat, l'initiative d'une proposition de loi visant à interdire les violences éducatives ordinaires revient à notre collègue Laurence Rossignol, qui interviendra tout à l'heure. Le Sénat a donc déjà adopté en mars dernier un texte excluant « les violences physiques ou psychologiques » de la pratique de l'autorité parentale. Je remercie notre collègue rapporteure, Marie-Pierre de la Gontrie, de nous proposer une synthèse en quelque sorte, une autre voie pour avancer de façon pragmatique et efficace. Sur le fond, l'interdiction des violences dites éducatives est un enjeu majeur de l'éducation de nos enfants. Il est aussi, n'en doutons pas, un moyen essentiel de changer le regard de notre société sur elle-même, de refuser que la violence puisse s'exprimer dans tout cadre, qu'elle puisse être tolérée et qu'elle relève de décisions individuelles ou de choix de vie. Élever les enfants dans la violence- leur parler fort, les menacer, les frapper, les humilier, les réprimer, les dénigrer systématiquement -, c'est dessiner trait à trait une société violente. Être violent devant ses enfants et vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est former des adultes à la violence, à être violents. Nous savons que nos enfants se construisent par mimétisme. Nous mesurons d'ailleurs la place qu'occupent les modèles parentaux dans la construction psychique des enfants. La docteure en psychologie clinique Karen Sadlier nous le rappelle. L'enfant confronté à des violences, dans le couple ou dans la famille, les banalise. Plus tard, il apprécie moins bien la peur et se met plus rapidement en danger et en fait un mode d'expression. Les pédiatres nous rappellent également que les traumatismes vécus dans l'enfance perdurent toute la vie, avec des conséquences psychologiques comme somatiques. Leur prise en charge représente un coût pour la société. Voilà pourquoi il faut que toute notre société en prenne conscience et agisse. Cette proposition de loi va dans le bon sens. Elle est nécessaire, mais évidemment pas suffisante : lorsque des situations de violence se font jour, elles doivent être signalées. Mes chers collègues, nous avons tous en tête une famille, une situation pour lesquelles nous nous demandons si l'enfant est vraiment bien traité, si la maladresse verbale, l'attitude des parents, leur perte de patience, leurs cris répétés nuisent pas à l'intérêt de l'enfant. Et puis, nous regardons ailleurs, la plupart du temps, même si nous en sommes très préoccupés. Dans ces situations de violences soupçonnées, je tiens à rappeler l'importance du signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes,

collègues, plutôt que de laisser une victime potentielle face aux auteurs de violences, même s'il s'agit de l'un de ses parents. J'en profite pour rappeler que le signalement est également essentiel chez tous les professionnels qui s'occupent d'enfants. Nous devons préciser le cadre législatif pour faire primer la protection de la victime sur l'exercice du secret professionnel.

Parce qu'être parent n'est pas du ressort de l'inné, parce que derrière un signalement, une aide va être apportée, nous devons signaler. Il y va de la protection des enfants et de la rupture du continuum des violences ; il y va surtout d'un autre regard de notre société sur les rapports

les violences subies par les enfants m'ont toujours interpellée. En tant qu'universitaire, ma thèse de droit portait sur le placement des enfants en souffrance intrafamiliale. Adjointe à la sécurité et à la prévention de Tourcoing, j'ai pu à maintes reprises constater que la frontière entre le tolérable et l'inadmissible des violences exercées sur les enfants par la famille était très fragile. Je me réjouis donc que ce sujet de l'interdiction des violences éducatives ordinaires soit débattu aujourd'hui dans notre Haute Assemblée. Je ne doute pas une seconde qu'une telle proposition de loi visant à les interdire sera aisément adoptée. Il y a de cela quelques décennies, il semblait normal de frapper ou d'humilier des enfants au sein des familles ou des établissements scolaires. certains de nos maîtres, considérant que nous étions trop bruyants- ou pas assez, au choix -, nous faisaient venir au tableau pour nous frapper le bout des doigts avec des règles en bois. D'autres, pour nous punir de bêtises d'enfants, avaient pris l'habitude de nous faire courir autour de la cour de l'école avec les mains sur la tête pour nous humilier aux yeux de tous. Je ne doute pas que vous vous en souveniez aussi, des années et des années après. Personne, à l'époque, n'y trouvait rien à redire et les parents doublaient souvent la punition au retour de l'écolier dans le foyer. C'était monnaie courante. Que de chemin parcouru ! Aucun parent aujourd'hui n'accepterait de telles violences « ordinaires » à l'école. Ces pratiques sont aujourd'hui considérées comme inadmissibles. Je m'en réjouis, comme vous tous, mais ne crions pas victoire trop vite : beaucoup de travail reste à faire, notamment pour faire cesser ces violences éducatives ordinaires dans les familles. Pourtant, la France s'est engagée depuis maintenant des décennies dans la protection de l'enfant. Les violences ordinaires peuvent prendre plusieurs formes psychologiques, lorsque l'enfant est victime de chantage, de menaces, de culpabilisations en tous genres ; physiques, lorsque l'enfant est victime de fessées, de gifles, de

ne permettent pas d'inculquer aux enfants un bon comportement, bien au contraire. C'est même l'inverse qui se produit. De nombreuses études ont en effet prouvé qu'un enfant exposé à des violences « ordinaires »- j'ai horreur de ce mot -a -a plus de chances de reproduire ce cercle vicieux en grandissant. La seule conclusion qu'il peut tirer de telles méthodes « éducatives », c'est que seule la violence de la loi du plus fort peut faire force de loi.

qui les pénaliseront dans leur vie future et dans leur rapport à l'autre. Le droit français interdit les violences envers les enfants dans son article 222-13 du code pénal et aggrave les sanctions lorsqu'elles sont commises par des ascendants légitimes. La France est signataire depuis 1990 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Et pourtant, ces violences subsistent. Cette proposition de loi qui vise à interdire les violences éducatives ordinaires est donc bel et bien d'actualité.

Alors, mettons tous les moyens en oeuvre pour que les violences ordinaires ne privent pas nos concitoyens les plus jeunes de ce temps si précieux pour leur épanouissement. Nous comptons sur vous tous, notamment sur vous, monsieur le secrétaire

mais nous ne laissons pas les enfants abandonnés sans aucune protection. Les lois sur la protection de l'enfance sont là, les services sociaux sont là et tous nos collègues élus dans des départements savent que nous agissons pour protéger nos enfants. Par ailleurs, je ne connais pas la différence entre la « vraie » violence et la « moindre » violence quand il s'agit d'enfants.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il est des « habitudes éducatives » qui font mal, au sens propre comme au sens figuré. Il est des coups, des brimades, des insultes qui semblent ne pas laisser de traces, mais qui peuvent faire des ravages. Tous les spécialistes et neuroscientifiques le confirment : fessées et « petites » gifles ne sont pas anodines pour la santé et le développement psychologique de nombreux enfants. Elles favorisent l'agressivité, fragilisent l'estime de soi, peuvent avoir une incidence sur les performances scolaires et compliquer la socialisation. Elles sont aussi, parfois, le terreau de châtiments plus graves. Par ce texte, il ne s'agit pas de se donner « bonne conscience », ni de multiplier les procureurs vertueux stigmatisant certains parents qui auront eu un geste regrettable ou une parole inappropriée. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre Le métier de parents est ô combien difficile. Les violences sont souvent synonymes de faiblesse, d'échec. Elles interviennent lorsqu'on n'a pas eu la patience, lorsqu'on n'a pas su trouver les mots. Mais il est aisé, confortablement installé dans ce bel hémicycle, de donner des leçons de morale, de prôner la pédagogie par l'explication, la compréhension, l'affection. Le coeur de cette proposition de loi, sa raison d'être, ce qu'elle peut et doit apporter, c'est une prise de conscience : la violence n'est jamais la solution, ce qui n'exclut pas la sanction. Depuis des années, certaines de nos collègues, d'Edwige Antier à Laurence Rossignol, ont mené ce combat, avec le succès relatif que l'on sait. Espérons que leur persévérance soit récompensée. Néanmoins,

il est une maltraitance sournoise, parfois plus dangereuse et plus destructrice : l'indifférence. Les coups sont condamnables, mais les silences s'ignorent. Certes, la loi ne peut pas tout. Mais toutes les graines de bienveillance qu'elle aura pu semer seront toujours des victoires et des progrès. Pour conclure, permettez-moi, monsieur le secrétaire d'État, de revenir sur votre double référence à Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau : il a peut-être bien écrit, mais il a bien mal agi ! L'auteur de l'a abandonné ses enfants ! Il n'est pas inutile de le rappeler. À chacun ses modèles et ses guides spirituels